L'ordre du jour appelle la désignation des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. En application de l'article 8, alinéa 3, de notre règlement, la liste des candidats présentés par les groupes a été publiée. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Les chiffres que je cite ici, mes chers collègues, visent à rappeler pourquoi nous avons déposé cette proposition de loi. Parce qu'elle résonne malheureusement avec l'actualité, car quand on touche 1 015 euros par mois, on doit souvent faire des choix entre payer ses factures, son loyer ou se nourrir. Notre proposition de loi ne tend pas à réduire, à elle seule, toutes les inégalités, mais elle vise à lutter contre la précarité énergétique, qui s'est accrue et pénalise celles et ceux qui sont déjà en grande difficulté.

Nous y sommes, et pourtant l'objectif est loin d'avoir été atteint. Les salaires et les pensions étant bloqués et le prix de l'énergie explosant, la situation s'est même dégradée.

Après les augmentations de plus de 7 % du tarif de l'électricité durant l'été dernier, c'est une nouvelle augmentation de 2,4 % qui pèse sur les ménages depuis le 1 février 2020. Et cela ne s'arrêtera pas de sitôt, puisqu'il est même annoncé que ces augmentations seront continues jusqu'en 2025 ! Or l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) indiquait que, avec 10 % d'augmentation- ce qui est déjà presque le cas cette année -, près de 420 000 ménages pourraient basculer en situation de précarité énergétique. Ainsi, après des mois de contestation des « gilets jaunes », des mobilisations toujours plus importantes contre la paupérisation comme seul horizon, voici votre réponse augmenter la facture d'électricité des particuliers de plus de 180 euros par an en moyenne en l'espace d'un an ! M. Carenco, le président la Commission de régulation de l'énergie affirmait il y a peu au Sénat que cette augmentation « n'est pas grave pour les ménages, car c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes par mois », ce qui confirme bien que certaines élites sont déconnectées de la réalité vécue par la majorité de nos concitoyens. Quel mépris phrase ! Contrairement à lui, nous affirmons que cette hausse aggrave les inégalités et fait basculer des dizaines de milliers de personnes en situation de précarité énergétique. Et contrairement à ce que le Gouvernement a affirmé, les usagers, devenus des clients, paient non pas le coût de l'énergie, mais bien le prix de l'Europe libérale. Ce sont 1,3 milliard d'euros pris dans les poches des ménages qui passent ainsi directement dans les coffres-forts des opérateurs privés avec les deux augmentations des neuf derniers mois. C'est donc un hold-up rondement mené au profit du privé, avec votre bénédiction. Avec ces différentes hausses, le peuple a compris une chose : le mythe selon lequel l'ouverture à la concurrence ferait baisser les prix est devenu une allégorie du mensonge. Depuis dix ans, l'électricité a augmenté de 27 % et le gaz de 70 %. Et pendant ce temps-là, vous préparez le démantèlement, la désintégration puis la future privatisation de l'entreprise publique avec le projet Hercule, à rebours du sens de l'Histoire, qui veut que seule une entreprise publique, intégrée et monopolistique puisse répondre aux défis d'avenir qu'est la transition énergétique et répondre aux besoins humains. Ces mêmes politiques de libéralisation plombent aujourd'hui EDF, l'obligeant à transférer à ses concurrents la rente du nucléaire sans contrepartie et sans engagement de leur part à investir. La hausse des tarifs réglementés intervient ainsi sur demande des opérateurs alternatifs privés à la CRE, afin qu'ils puissent proposer des tarifs libres au même prix que les tarifs réglementés. Tout cela, au final, pour respecter le dogme de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée imposé par Bruxelles, même lorsque cette concurrence est défaillante. Alors que la solution adoptée consiste à confier Alors que la solution adoptée consiste à confier la régulation des prix au marché, méthode inefficace s'il fallait encore le démontrer, notre proposition de loi choisit de consacrer l'accès à l'énergie en droit fondamental, tel que garanti par la Constitution, gardienne de notre histoire et des droits fondamentaux qui en ont émergé. Sous la monarchie absolue sont nées les revendications de libertés citoyennes et politiques. Avec la révolution industrielle, les premières garanties économiques et sociales ont été conquises, enrichies par le Front populaire et le Conseil national de la Résistance. Ce sont ensuite les catastrophes écologiques et la prise de conscience du danger futur qu'elles supposent qui ont introduit l'impératif de droits collectifs et de protection de l'environnement. Alors que nous combattons sans relâche pour préserver et enrichir ces droits conquis de longue date, il nous faut inclure dans ces luttes la création de droits nouveaux. Ériger l'accès à l'énergie en droit fondamental, comme nous le proposons à l'article 1, s'impose comme une suite logique à cette dynamique historique qui fait correspondre nos droits fondamentaux aux nécessités de notre temps. Il s'agirait également de respecter nos engagements en donnant un fondement national aux dispositions du socle des droits sociaux de Göteborg, lequel place l'énergie parmi les services essentiels auxquels toute personne a le droit d'accéder. Oui, nous le disons : alors que les différents gouvernements, prônant une politique libérale, essaient de réduire depuis trente ans les droits et les accès aux droits, nous prônons une vision de la société radicalement différente. Nous voulons la garantie d'accès aux droits et en conquérir de nouveaux. Si nous votons ce premier article, il conviendra donc ensuite de garantir l'accès à ce droit. Cet objectif d'égalité dans l'accès à l'énergie doit s'accompagner de celui de justice sociale. Nous voulons, à travers l'article 2, que soient interdites tout au long de l'année les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz. Et ainsi, en finir avec ce scandale consistant à priver des hommes et des femmes d'électricité et de gaz, c'est-à-dire pouvoir se doucher, se chauffer ou encore manger. Il y a quelques jours, à la suite d'actions syndicales des syndicalistes de l'énergie ont coupé quelques instants l'électricité dans des lieux symboliques pour faire entendre leur voix contre la réforme des retraites, nous avons entendu la droite sénatoriale et le Gouvernement pousser de concert des cris d'orfraie et demander des sanctions exemplaires. Mais, bizarrement, personne n'a fait part de sa vive émotion lorsque, l'an dernier, 574 000 ménages ont vu leur électricité coupée ou réduite. Car, oui, en France, une entreprise, publique ou privée, peut punir les pauvres, parce qu'ils sont pauvres. Nous disons aux syndicalistes que vous accusez de tous les maux, qui sont les mêmes que ceux qui rétablissent le courant en se nommant les Robins des Bois et qui sont poursuivis pour délit de solidarité, que nous les soutenons pleinement. Enfin, nous entendons sortir l'énergie du secteur marchand pour lui reconnaître le statut de bien de première nécessité, afin d'y appliquer, via notre article 4, et en vertu de la directive du Conseil européen du 19 octobre 1992, un taux réduit de TVA à hauteur de 5,5 %. Cette mesure d'allégement fiscal prend tout son sens lorsque l'on se livre à un examen de la composition du prix de l'électricité. Les taxes pèsent pour un tiers dans la facture payée par les usagers, ce qui est déjà lourd de conséquences financières pour les ménages précaires et rend la facture illisible. En l'état, cela veut dire toujours plus de vulnérabilité pour les 7 millions de ménages qui se trouvent en situation de précarité énergétique. Enfin, après l'allégement de la TVA à 5,5 %, nous proposons que les bénéficiaires du chèque énergie soient exonérés de taxes sur la consommation d'électricité et de gaz, et à raison (CSPE), censée financer les énergies renouvelables, demeure un dispositif à la gestion et aux résultats opaques. Elle est aujourd'hui absorbée directement dans le budget de l'État et a donc servi par exemple à financer le

La commission n'a pas adopté notre proposition de loi et propose de travailler sur le chèque énergie. Nous rappelons que cette solution curative n'est pas durable et qu'en plus il faudrait, selon l'Agence de l'environnement et

car ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Mais nous pensons surtout que la majorité des personnes concernées veulent non pas recevoir l'aumône, mais plutôt pouvoir payer leur facture. Il est donc urgent d'augmenter les salaires. salaires. Évidemment, cette proposition de loi ne répondra pas seule à la question de la précarité énergétique. Il faut mettre en place des politiques publiques ciblées sur les facteurs qui fragilisent les ménages- revenu disponible, prix de l'énergie, conditions de vie, qualité de l'habitat et de l'équipement de chauffage. On est d'accord ! Ce dernier point est important. Nous le redisons, comme nous l'avons affirmé pendant l'examen de la loi ÉLAN : il faut d'urgence un plan Marshall de la rénovation énergétique des logements. Au rythme actuel, il faudrait cent quarante ans pour rénover l'ensemble des logements classés F et G. Les aides existantes sont par ailleurs aujourd'hui majoritairement destinées aux propriétaires, alors que la grande majorité des ménages précaires demeurent locataires. Il faut vraiment conclure. Cette proposition de loi est donc un pas

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous mesurons tous, dans notre vie quotidienne, l'importance de disposer d'une énergie en quantité suffisante et à un prix raisonnable. Sans énergie, il est impossible de se chauffer, de se déplacer, voire de communiquer ou de s'informer. C'est donc un poste essentiel dans le budget des ménages et une dépense contrainte qu'il est souvent difficile de maîtriser,

près de 6,8 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique au sens économique, c'est-à-dire que sont concernés les ménages pauvres et modestes consacrant plus de 8 % de leurs revenus au paiement de la facture énergétique de leur logement. La question abordée par la proposition de loi de nos collègues du groupe communiste est donc majeure et chacun partage, à l'évidence, la préoccupation exprimée par ses auteurs pour faciliter l'accès à l'énergie ou réduire la facture- j'oserai dire : la fracture énergétique. Pour autant, la commission a jugé qu'aucune des mesures proposées par le texte n'était satisfaisante et que d'autres pistes devaient être explorées pour répondre à ces enjeux, j'y reviendrai. En premier lieu, nos collègues proposent d'élever l'accès à l'énergie au rang de droit fondamental. Comme tous nos interlocuteurs l'ont confirmé, cette mesure n'aurait, en elle-même, aucun effet juridique notable ; elle ne changerait rien sur le plan fiscal, pas plus qu'elle n'octroierait, à elle seule, de nouveaux droits. La deuxième mesure proposée serait, quant à elle, bien concrète. Elle consisterait à étendre l'interdiction des coupures d'électricité, de chaleur et de gaz, qui ne vaut aujourd'hui que durant la trêve hivernale, à l'ensemble de l'année, comme c'est déjà le cas pour l'eau. Cette protection nouvelle serait accordée uniquement aux bénéficiaires du chèque énergie. de nombreux motifs nous ont conduits à écarter cette solution. Elle reviendrait d'abord à déresponsabiliser une partie des usagers et augmenterait immanquablement les impayés, dont le coût se reporterait sur l'ensemble des consommateurs, y compris les plus modestes. Le retour d'expérience de l'eau le démontre : dans les trois années suivant l'interdiction des coupures tout au long de l'année, les impayés et irrécouvrables ont augmenté de 20 %, selon les données de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Ensuite, elle tendrait aussi à masquer le coût réel de l'énergie et n'inciterait pas à la maîtrise des consommations, ce qui irait à l'encontre de nos objectifs climatiques. Cette mesure, qui est adossée au dispositif du chèque énergie, poserait par ailleurs des difficultés en termes d'identification des bénéficiaires pour les fournisseurs, en particulier lorsque le chèque énergie a été affecté par leur client à un autre fournisseur. Elle pourrait ainsi conduire à des effets d'aubaine importants si, du fait de ces difficultés d'identification, et pour éviter tout risque de contentieux, elle venait à protéger indifféremment les ménages précaires et les ménages solvables. À l'inverse, certains publics précaires n'en bénéficieraient pas, car l'ensemble des ménages n'est pas éligible au chèque énergie. Il en est ainsi des personnes en réinsertion vivant dans des logements en intermédiation locative. Enfin, il faut rappeler que, si tout doit être fait, bien sûr, pour éviter sa mise en oeuvre effective, l'annonce d'une possible coupure déclenche le plus souvent un processus d'évaluation de la situation du consommateur, d'orientation vers les différentes aides disponibles et d'étalement des paiements qui permet, bien souvent, de sortir de cette spirale d'accumulation de dettes. Les deux autres mesures proposées visent le même objectif : celui d'alléger la facture en modulant le niveau de la fiscalité énergétique, mais selon des modalités bien différentes.

; la seconde mesure proposée établirait un taux réduit de TVA à 5,5 % sur une partie des consommations, dont le niveau serait fonction, notamment, de la composition familiale du foyer, mais sans condition de ressources. Là aussi, nous pouvons partager le constat- celui de la hausse des taxes sur l'énergie au cours des dernières années - de même que l'objectif- celui d'alléger la facture des Français mais sans pour autant partager les solutions préconisées, qui seraient à la fois complexes, sinon impossibles à mettre à oeuvre, et largement inefficaces sur le fond. Sur le plan juridique d'abord, le droit européen n'autorise pas l'application de régimes d'exonération ou de taux différents entre les ménages. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que l'on ne peut pas faire de redistribution au profit des ménages les plus modestes, mais alors il faut passer par des outils plus adaptés, à commencer par des aides directes. Sur le plan pratique, ensuite, ces mesures rendraient plus complexe la facturation, avec des risques d'erreurs et des surcoûts importants, et les fournisseurs devraient même, pour appliquer la mesure sur la TVA, connaître la composition du foyer à chaque période de facturation, ce qui poserait clairement question en termes de protection de la vie privée. Enfin, le rapport coût-efficacité de ces mesures serait très peu favorable selon nos calculs : la perte de recettes pour l'État serait d'au moins 2,5 milliards d'euros par an pour une mesure qui bénéficierait, dans le cas de la TVA, à tous les consommateurs, y compris ceux qui peuvent s'acquitter de leur facture sans difficulté particulière. Il me semble que nous pourrions trouver un meilleur usage de ces montants pour cibler, en priorité, les plus modestes. Pour ce faire, notre commission préconise d'améliorer et d'amplifier les dispositifs existants. Lesquels ? Tout d'abord, il importe de réduire le taux de non-recours au chèque énergie, qui demeure important puisqu'il s'établirait à ce jour entre 20 % et 25 %. En effet, de multiples retours de terrain de la part de travailleurs sociaux, d'élus locaux, d'associations font encore état de difficultés à appréhender le dispositif. Deux leviers peuvent corriger cela : d'abord, intensifier la communication sur le chèque énergie, pour que l'information parvienne bien à tous ses bénéficiaires potentiels parallèlement, il convient de simplifier son fonctionnement autant que possible, madame la secrétaire d'État, pour que ceux qui y ont droit ne se censurent pas par « phobie administrative Au demeurant, il faudrait également augmenter les montants maximaux du chèque énergie pour les tranches de revenus les plus basses. Durant l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté une hausse des crédits alloués au chèque énergie de 75 millions d'euros, soit en moyenne 25 euros par ménage, contre l'avis du Gouvernement.

du revenu des ménages les plus modestes. Certes, le barème du chèque énergie a été augmenté en 2019, et je salue cette initiative, mais cette évolution reste insuffisante pour permettre à ces ménages de régler leurs factures, sans parler de couvrir leurs frais de rénovation énergétique. Plus généralement, la précarité énergétique est un mal qu'on ne pourra éradiquer seulement en octroyant des aides au paiement des factures d'énergie. Ces mesures, telles que le chèque énergie, sont évidemment essentielles pour faire face à l'urgence, mais elles ne font que traiter les symptômes de la précarité énergétique. Pour réduire celle-ci, il est aussi nécessaire d'amplifier la politique de rénovation énergétique des logements en continuant les efforts de simplification des dispositifs d'aides entamés en ce début d'année par le Gouvernement, sans renier pour autant leur niveau d'ambition. Je pense notamment au lancement de la prime unifiée MaPrimeRénov'. Enfin, d'autres mesures pourraient être envisagées : par exemple sanctionner les fournisseurs qui ne respectent pas l'interdiction de rattrapage des factures de plus de quatorze rendre obligatoire la contribution de l'ensemble des fournisseurs au fonds de solidarité pour le logement, ou encore étendre l'interdiction des coupures durant la trêve hivernale au gaz

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, les mesures de lutte contre la précarité énergétique figurant dans cette proposition de loi abordent un vrai enjeu de politique publique. La précarité énergétique est une réalité forte pour nombre de nos concitoyens. C'est un enjeu de transition énergétique et de lutte contre la pauvreté et le Gouvernement travaille pour y apporter des solutions. L'ONPE, que vous avez cité, définit la précarité énergétique comme « le fait de consacrer plus de 8 % de ses revenus au paiement des factures d'énergie du logement En 2018, 11,7 % des Français étaient au-dessus de ce seuil, contre 14,5 % en 2013. Les progrès sont donc réels, mais, je le reconnais tout à fait, trop lents. Au-delà des chiffres, la précarité énergétique est d'abord une réalité de difficultés individuelles, de ménages qui vivent dans un logement inconfortable, pour qui les dépenses de chauffage et de transport sont élevées, qui ont du mal à payer leurs factures. En 2017, 123 000 ménages ont bénéficié d'une aide des fonds de solidarité pour le logement pour payer leurs factures d'énergie. En 2018, 572 000 interventions des fournisseurs d'énergie ont eu lieu à la suite d'impayés, c'est-à-dire des réductions de puissance, des suspensions de fourniture ou même des résiliations de contrat. Si ce nombre était de 624 000 en 2014, il montre bien l'ampleur du phénomène. Nos concitoyens nous ont rappelé ces difficultés au cours des derniers mois. Ils nous ont dit que la fluctuation des prix de l'énergie avait sur eux un impact important. La proposition de loi que vous présentez aujourd'hui a donc retenu toute l'attention du Gouvernement. Néanmoins, si son objectif, auquel nous souscrivons, est louable, les moyens qu'elle propose pour y parvenir ne nous semblent pas les mieux adaptés. En effet, la proposition de loi entre en désaccord direct avec plusieurs engagements européens de la France, notamment en termes d'encadrement de la fiscalité. Il est ainsi impossible, en matière de fiscalité de l'énergie, d'opérer une distinction entre les ménages en fonction de leurs revenus, Le soutien à ces ménages peut en revanche passer par d'autres moyens, comme ceux que le Gouvernement a mis en oeuvre et continuera à soutenir, par exemple le chèque énergie. En outre, En outre, seule la Constitution peut élever un principe au rang de droit fondamental. La loi ordinaire n'est pas un vecteur suffisant, d'autant plus que l'électricité est d'ores et déjà considérée par les tribunaux comme un bien de première nécessité. Enfin, la Enfin, la Commission de régulation de l'énergie suit en permanence la situation du marché de l'énergie, pour le gaz naturel comme pour l'électricité. Elle produit à ce sujet une documentation riche et abondante. Pour cette raison, il nous semble donc peu utile de présenter un rapport supplémentaire, qui ne viendrait pour l'essentiel que répéter ce que d'autres disent déjà. Le Gouvernement est à l'écoute de ces difficultés et souhaite être force de propositions. C'est pourquoi, au-delà des dispositifs déjà en place, nous avons, depuis 2017, renforcé les mesures de lutte contre la précarité énergétique. Les coupures d'électricité et de gaz naturel étaient déjà interdites pendant la trêve hivernale afin de protéger tous les ménages ; mais, au-delà de l'interdiction de coupure, des protections supplémentaires sont mises en oeuvre pour les bénéficiaires du chèque énergie sur leurs contrats d'électricité et de gaz naturel. Ainsi, en cas d'incident de paiement, ces ménages bénéficient du maintien de leur puissance électrique pendant l'hiver, d'une réduction des frais liés à une intervention en cas d'impayés et d'une exonération des frais liés à un rejet de paiement. De plus, dans le cas où un fournisseur envisagerait de mettre en oeuvre une coupure, il est important de rappeler que les pratiques des fournisseurs sont très encadrées. En effet, l'annonce d'une possible coupure ou d'une réduction de puissance déclenche un processus d'évaluation de la situation du client, d'orientation vers les aides disponibles et d'étalement des paiements. En ce sens, elle fait office de signal d'alerte et permet de déclencher un processus d'accompagnement pour aider le consommateur en difficulté. Par ailleurs, pour accompagner financièrement les ménages, le chèque énergie, créé sous forme expérimentale par la loi de 2015, a été généralisé en 2018, année où il a été ouvert à plus de 3,6 millions de ménages. Disponible quel que soit le mode de chauffage, ce dispositif est plus efficace que les anciens tarifs sociaux, limités à l'électricité et au gaz. En 2019, afin d'améliorer l'accompagnement des ménages précaires, le Gouvernement a élargi le chèque énergie chèque énergie à 5,7 millions de ménages et augmenté de 50 euros les montants versés par rapport à 2018. Près de 850 millions d'euros sont désormais consacrés à cette aide. Ce chèque énergie est en train de trouver son public. Le taux de recours s'est établi à environ 80 % en 2018 ; il sera supérieur en 2019 et le Gouvernement travaille à la simplification des des formulaires, des messages d'information, à l'automatisation du versement, pour augmenter encore ce taux de recours au-delà du montant un peu supérieur à 80 % auquel il va se situer cette année. cette année. Notre effort doit aussi se concentrer sur les sources du problème et nous devons réduire directement et sur le long terme le poids des factures d'énergie. C'est la raison pour laquelle nous menons une politique ambitieuse en matière de rénovation de logements. Le Gouvernement vise un objectif de 500 000 rénovations énergétiques par an, dont 150 000 au titre des passoires énergétiques qui sont généralement occupées par les ménages les plus fragiles. C'est insuffisant ! Cela inclut également 100 000 rénovations par an de logements sociaux.

Je pense aussi à la mobilisation des certificats d'économies d'énergie, notamment les « Coups de pouce ». Ces certificats d'économies d'énergie apportent des moyens importants, en finançant des investissements et en soutenant des programmes de détection et d'accompagnement des ménages. Ces dernières années, les certificats d'économies d'énergie dits « de précarité énergétique » ont représenté un financement d'environ un milliard d'euros par an. En 2019, le Gouvernement a modifié le dispositif « Coup de pouce économies d'énergie » financé par les certificats d'économies d'énergie à renforcer très fortement les aides pour les changements de moyens de chauffage et les travaux d'isolation. Ces évolutions ont eu un fort effet d'entraînement, en particulier pour les ménages modestes, pour lesquels ces coups de pouce sont bonifiés

Grâce aux mesures sur l'isolation, les économies sont estimées à environ 300 millions d'euros sur les factures et 700 tonnes de CO2 évitées. Enfin, l'éco-prêt à taux zéro a été fortement simplifié en 2019 : il peut désormais assurer le financement d'un seul geste de rénovation sans notion de bouquet de travaux.

laquelle nous souhaitons des adhésions les plus larges possible. Cette charte est aujourd'hui signée par plus d'une centaine d'acteurs et nous avons proposé aux collectivités locales, notamment aux régions, aux départements et aux de s'engager avec nous sur la pérennisation et l'amélioration des plateformes d'information et de conseil à travers un programme de certificat d'économies d'énergie qui permet de financer ces plateformes à hauteur de 200 millions d'euros pour les trois prochaines années. Le débat d'aujourd'hui nous invite à aller encore plus loin. C'est ce que nous allons faire. Sur la rénovation des bâtiments, il nous faut à la fois rendre nos dispositifs de soutien encore plus efficaces dans leur conception et plus ciblés vers nos concitoyens les plus fragiles, en renforçant la détection et l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. Pour 2021, nous finirons la transformation du CITE en prime

Nous continuerons à mobiliser les programmes de certificats d'économies d'énergie pour tester des innovations qui visent à réduire le coût des rénovations et à les généraliser. À titre d'exemple, le dispositif continuera à soutenir le déploiement en France du programme EnergieSprong dans les logements sociaux, mais aussi dans le parc privé et les bâtiments éducatifs.

elle fixe l'exigence d'une performance énergétique minimale à respecter à partir du 1 janvier 2023 pour que le logement puisse être qualifié de décent, et donc mis en location. Avant 2028, les propriétaires de passoires thermiques devront avoir réalisé des travaux d'amélioration de la performance énergétique permettant à leur logement d'atteindre au moins la classe E. La loi relative à l'énergie et au climat doit ainsi conduire à l'éradication des logements de classe F et G d'ici au 1 janvier 2028 pour les maisons individuelles et la plupart des copropriétés et d'ici au 1 janvier 2033 pour les copropriétés confrontées à des difficultés particulières. Ces mesures et obligations seront rendues possibles en prenant appui sur le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) qui, grâce à une concertation et un travail avec les professionnels, sera amélioré pour le rendre fiable et opposable en 2021. La première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui court jusqu'en 2023, permettra d'analyser plus finement la composition du parc de logements et de mieux connaître les propriétaires de passoires thermiques. À la lumière de ces études et des résultats obtenus durant la phase d'incitation, des sanctions en cas de non-respect des obligations de travaux d'ici à 2028 pourront être définies en 2023 dans le cadre de la loi de programmation quinquennale sur l'énergie. En conclusion, j'aimerais réaffirmer l'engagement du Gouvernement : les ménages les plus vulnérables ne doivent pas être laissés sur le côté et la transition écologique doit être également solidaire. Ces actions concrètes et les projets pour les prochains mois montrent que le soutien aux plus vulnérables est au coeur de nos préoccupations et de nos actions. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, bien que louable dans son objectif, ne me semble pas la meilleure manière de lutter contre la précarité énergétique. Le désaccord avec cette proposition de loi ne signifie pas que nous ne partageons pas ses objectifs ; il signifie simplement que nous proposons d'autres moyens, plus efficaces, pour concilier allégement des factures des plus vulnérables et incitation au changement des comportements.

Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que nous avons adopté dans le cadre de la loi relative à l'énergie et au climat, chacun doit disposer des moyens de réaliser concrètement la transition énergétique. Or la précarité énergétique est un phénomène en hausse

C'est pourquoi nous devons être très attentifs au poids de l'énergie dans le portefeuille des Français : sur ce point, rappelons que la fiscalité énergétique atteint 3 000 euros par an et par ménage, jusqu'à 4 000 euros en zone rurale, et que le transport et l'énergie représentent

l'objectif de lutte contre la précarité énergétique visé par la présente proposition de loi, les évolutions qu'elle emporte ne sont pas satisfaisantes. En premier lieu, la consécration de l'énergie comme un droit fondamental présente un caractère largement incantatoire. Ensuite, l'application tout au long de l'année de la trêve hivernale comporte un effet d'aubaine évident sans apporter de véritable fond. En outre, les réductions de TVA, de CSPE et de TICGN ne sont pas conformes au droit européen qui prohibe la différenciation des taux selon la situation des ménages. Enfin, la demande de rapport apparaît comme une réponse bien modeste au regard de la gravité des enjeux. Pour autant, la question qui est posée est très

ne sert donc à rien ! Cette loi a en outre renforcé les informations que les fournisseurs d'électricité et de gaz doivent transmettre à plusieurs instances de régulation, ce qui concourt à la protection des consommateurs.

l'initiative de sa commission des affaires économiques, suivait une recommandation du médiateur national de l'énergie. Je déplore aussi que les mesures concrètes que j'avais défendues avec mes collègues Jean-François Husson et Dominique Estrosi Sassone aient connu le même sort ; je veux parler ici des coups de pouce proposés dans le cadre de la réforme du CITE pour le renouvellement par les ménages modestes d'équipements du quotidien. Nous considérons que les moyens déployés par le Gouvernement doivent être rehaussés à la hauteur des objectifs votés par le législateur. Comment atteindre l'objectif fixé dans la loi relative

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comment un pays comme la France peut-il laisser des enfants et des adultes souffrir du froid dans leur logement ? N'est-il pas temps de revenir aux principes d'une économie morale et de travailler à la formulation d'un droit à une existence digne ? Cette proposition de loi du groupe CRCE va dans le bon sens et, au nom du groupe socialiste, j'indique ici que nous la soutenons. Personne n'échappera aux conséquences des bouleversements climatiques, de la dégradation de la qualité de l'eau et de l'air ou de l'effondrement de la biodiversité, mais les plus touchés, et de loin, seront les plus pauvres, alors qu'ils sont les moins responsables de la situation. Ce sont eux, d'ailleurs, qui habitent les logements les plus insalubres. Ce sont eux qui vivent dans des passoires énergétiques, dont les propriétaires récalcitrants s'opposent à la réalisation de travaux de rénovation thermique. Le mal est trop grave pour que l'on tergiverse, encore, ou que l'on reporte les décisions. Ce n'est pourtant pas faute d'entendre les alertes lancées par la Fondation Abbé Pierre, selon laquelle il est plus que temps de changer de dimension, ou celles de l'Observatoire des inégalités qui regrette que la lutte contre la pauvreté ne soit pas à la hauteur des enjeux sociaux. On sait que l'année 2019 a été celle d'un triste record, celui du nombre de coupures d'énergie pour impayés. Les trois facteurs de la précarité énergétique sont connus

Notez que le prix de l'électricité a augmenté de 40 % en dix ans, que la CSPE a été multipliée par cinq, que les taxes pèsent à hauteur de 35 % sur le prix de l'électricité, de 27 % sur celui du gaz, et que la TICGN a été multipliée par

Nul ne conteste que des efforts aient été réalisés au cours de ces dernières années pour lutter contre la précarité énergétique, mais ces efforts ne sont pas à la hauteur des enjeux sociaux. C'est aussi l'ONPE qui précisait que, pour sortir l'ensemble des ménages de la précarité énergétique, l'aide nécessaire s'élèverait à 3 milliards d'euros par an. En fait, pour que le taux d'effort soit inférieur à 8 % des revenus, l'aide par logement devrait être de l'ordre de 710 euros par an.

Il s'agit par exemple de la question des rattrapages de facturation portant sur des périodes assez longues. La loi relative à la transition énergétique de 2015 prévoit que les fournisseurs d'électricité et de gaz n'ont pas le droit de facturer des consommations intervenues plus de quatorze mois avant le dernier relevé de compteur.

Cela dit, nous soutenons, avec le même souci de lutter contre la précarité énergétique, les mesures proposées par Fabien Gay et son groupe. Ainsi, la proposition de loi prévoit d'élever l'accès à l'énergie au rang de droit fondamental. Je rappelle que l'énergie est reconnue comme un bien de première nécessité. Comme cela est précisé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'accès à l'énergie et à l'électricité en particulier est devenu une nécessité qui ne se limite pas au chauffage durant la période hivernale. Pour éviter l'exclusion, l'accès à l'énergie est une impérieuse

aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité ». Certes, j'ai bien noté que certains d'entre nous émettent des doutes quant à la portée normative d'une telle mesure, mais je relève également que l'on n'écarte pas l'idée- je cite Mme le rapporteur -qu'elle pourrait donner une plus grande chance de succès aux procédures de référé, voire entraîner l'automaticité de certains dispositifs- aide juridique systématique, fournisseur de dernier recours ... -et ouvrir la voie à

précarité énergétique, il s'agit d'une mesure cohérente avec la précédente. C'est une protection supplémentaire pour les plus fragiles. Je m'étonne que l'on nous parle encore d'effet d'aubaine, d'autant que je me souviens que, lorsque nous avons instauré l'interdiction des coupures d'énergie durant l'hiver,

nous partageons le souci du groupe CRCE d'exonérer de la TICGN et de la CSPE les ménages précaires, car force est de constater que la fiscalité de l'énergie n'est pas étrangère aux difficultés financières de certains ménages, ces les faisant basculer dans la précarité énergétique. Concernant l'article 4, et pour les mêmes raisons que précédemment, nous proposerons un amendement visant à élargir le périmètre du taux réduit de TVA à une première tranche de consommation d'énergie dite de première nécessité, mais pour les seuls bénéficiaires du chèque énergie. En effet, un taux de TVA de 20 % est très pénalisant

Cette double taxation n'est pas acceptable pour ceux qui sont dans la difficulté et qui se chauffent au fioul, à l'électricité ou au gaz. Enfin, je pense serait intéressant que soit effectué un bilan de la libéralisation du marché de l'énergie. Si, depuis 1960, les prix de l'électricité sont inférieurs en France à ceux de nos voisins européens, nous le devons à notre mix énergétique et aux tarifs réglementés.

trop cédé sur ce terrain et il ne faudrait pas remettre en cause ce qui reste des tarifs réglementés. Selon les propos tenus en mai dernier par le médiateur de l'énergie, la concurrence n'a pas fait baisser les prix ; ils ne pouvaient qu'augmenter en raison des besoins de financement des énergies renouvelables, prix de revient du nucléaire en hausse du fait du grand carénage et de la construction de l'EPR, etc. Mais le médiateur ajoutait que la séparation des activités de fourniture et de distribution, rendue nécessaire par l'ouverture des marchés, donc par la libéralisation, a conduit à une « désoptimisation » des organisations, et donc à des coûts additionnels, notamment en matière de systèmes d'information. Par ailleurs, je relève que, si 39 % des Français estiment que la multiplication des fournisseurs va permettre de faire jouer la concurrence, ils sont presque autant à estimer que cela aboutit à une jungle d'offres peu lisibles, à des risques d'abus et de dérives, à une qualité de service dégradée et à des prix en hausse ou fluctuants. Je note que 86 % des Français apprécient les tarifs réglementés qui assurent stabilité, sécurité et cohésion territoriale et sociale et qui sont aussi un point de repère pour les consommateurs qui hésitent à opter pour une offre de marché. Cela dit, si l'urgence consiste à aider les personnes en situation de précarité à payer leurs factures, la meilleure manière d'agir

trop lointaines et, pour l'heure, le reste à charge est trop élevé. En fait, dans le contexte climatique actuel, l'objectif est bien de faire reculer la précarité énergétique, tout en oeuvrant pour une société plus respectueuse des ressources naturelles. Dès lors, le principal levier pour lutter contre la précarité est la rénovation thermique des logements. Éradiquer les logements passoires, c'est résoudre en grande partie la précarité énergétique. Problème : trop de propriétaires sont récalcitrants ou ignorent les possibilités d'aides. Pour conclure, je dirai que, depuis des années, nous pensons tous ici que l'urgence commande de faire disparaître la précarité énergétique. Nous avons aujourd'hui la possibilité de mettre en accord nos actes avec nos discours. Ne nous contentons pas de dénoncer ce problème ! Combattons-le en pensant que rien, jamais, ne doit contrevenir à un principe aussi simple que fondamental, celui du droit à une existence digne. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, facteur déclenchant de la crise des « gilets jaunes », l'augmentation du prix de l'énergie amplifiée par l'application de diverses taxes sur une même assiette demeure peu intelligible et peu acceptable pour nos concitoyens. Le gel des tarifs de l'électricité et du gaz annoncé en janvier 2019 par le Premier ministre lui avait permis de lâcher du lest, le temps de l'hiver. L'extension du bénéfice du chèque énergie de 3,6 millions à 5,8 millions de personnes a de plus redonné du pouvoir d'achat à ceux qui en avaient le plus besoin. Toutefois, ces mesures sont insuffisantes pour lutter contre la précarité énergétique qui concernait encore 6,7 millions de personnes en 2017. Or celles-ci consacrent plus de 8 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Mes chers collègues, souscrivons aux objectifs de la présente proposition de loi et je remercie Fabien Gay et le groupe CRCE de cette initiative, tout en considérant que les mesures proposées ne sont pas les plus pertinentes pour instaurer un droit effectif à l'accès à l'énergie lutter contre la précarité énergétique. Cependant, la majorité de notre groupe ne peut pas souscrire aux deux principales dispositions de ce texte, à savoir l'interdiction des coupures en matière d'énergie et les exonérations fiscales prévues. Sur l'interdiction des coupures d'électricité, de chaleur et de gaz tout au long de l'année, nous craignons qu'elle ne profite davantage aux mauvais payeurs qu'aux ménages en difficulté qui sont les premiers à honorer leurs dettes. La majorité du groupe du RDSE ne soutiendra donc pas ce que nous considérons comme une manière de déresponsabiliser les consommateurs, alors que le droit en vigueur est suffisamment équilibré. Cela a été dit, les coupures restent interdites au cours de la trêve hivernale, période où la consommation est au maximum et la dépense la plus contrainte. En outre, des délais supplémentaires sont accordés en cas de non-paiement de la facture,

Mais encore faudrait-il que les ménages en situation de précarité connaissent les dispositifs d'aide. Il est d'ailleurs préférable d'en accroître la lisibilité et, surtout, de les affecter aux plus fragiles- Mme la rapporteure À ce titre, l'introduction du chèque énergie devrait permettre de réduire le taux de non-recours. Renforçons donc l'existant et consacrons davantage de moyens à la rénovation du bâti. Pour l'ensemble de nos concitoyens, le logement est la première dépense contrainte, sans oublier bien sûr le surcoût des passoires thermiques. Le saupoudrage des subventions publiques nuit à leur efficacité. La remise à plat déjà engagée des aides va dans le bon sens. les mesures fiscales, outre leur non-conformité au droit européen et leur coût élevé pour nos finances publiques après les mesures prises par le Gouvernement en matière de pouvoir d'achat, nous sommes une nouvelle fois de l'avis de notre rapporteure sur l'inapplicabilité de l'exonération de TICGN et de CSPE des ménages éligibles au chèque énergie, puisqu'il faudrait que le fournisseur ait connaissance à tout moment du statut du ménage. De même, la mise en oeuvre opérationnelle du taux de TVA réduit applicable à la première tranche de consommation d'énergie, « en tenant compte notamment de la situation familiale », est pour le moins douteuse. Cela m'évoque un souvenir, celui de la tarification progressive de l'énergie, principale disposition de la proposition de loi Brottes avant qu'elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel ... Idée intéressante par sa dimension à la fois sociale et environnementale, elle instaurait dans les faits une usine à gaz, raison pour laquelle j'avais voté la suppression de cet article. Enfin, il faut rappeler que la taxation élevée qui pèse sur l'énergie n'est pas une spécificité française. Peut-être faudrait-il avant tout simplifier la facture énergétique ? Et surtout, comme nos concitoyens l'exigent, faire en sorte que la fiscalité écologique soit affectée à la transition énergétique. Mes chers collègues, l'énergie a un coût, ce qui permet d'inciter à la sobriété et à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Cela ne veut pas dire pour autant que nous justifions l'augmentation continue des tarifs de l'électricité. Le coût de l'énergie fait l'objet d'un mode de calcul précis reposant sur une base légale afin de protéger les consommateurs et de les faire bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire. N'oublions pas les avantages attendus de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité,

Or la France se caractérise par la multiplication récente de fournisseurs qui ne produisent pas d'électricité et qui parviennent à se différencier de l'opérateur historique par leurs services et leurs offres d'électricité, même si celle-ci La délibération de la CRE proposant une augmentation de 5,9 % des tarifs réglementés de vente d'électricité a été contestée par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 25 mars 2019. La loi relative à l'énergie et au climat offre la possibilité de relever le plafond du tarif à laquelle le Gouvernement n'a pas eu recours. Il faudra donc éviter à l'avenir de maintenir l'ouverture à marche forcée à une concurrence artificielle au détriment du consommateur. Cela n'est conforme ni aux principes généraux du droit de la concurrence ni aux objectifs de l'ouverture du marché européen de l'énergie. Comme l'a affirmé le Conseil d'État dans sa décision du 18 mai 2018, l'électricité est un produit de première nécessité non substituable. C'est ce statut particulier qui nous permet de préserver les tarifs réglementés de vente, contrairement à ce qui a été décidé pour le gaz. Nous serons donc particulièrement vigilants, lors de la prochaine réforme portant nouvelle régulation économique du nucléaire existant, à ce que les consommateurs ne soient pas les perdants de l'ouverture à la concurrence. Dans cette attente, la majorité des membres du groupe du RDSE s'abstiendra

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce matin a trait à la précarité énergétique et, plus globalement, à l'accès de tous à l'énergie, sujet plus que prégnant dans la France d'aujourd'hui. Pour les ménages les plus modestes, la part du budget consacrée aux dépenses d'énergie, en particulier au chauffage, devient une charge importante, parfois insurmontable. L'énergie est en effet indispensable pour se chauffer et pour se déplacer, mais aussi pour de nombreux actes de la vie quotidienne, tout en étant une dépense contrainte qui, bien souvent, mobilise une part importante du budget des ménages. Pour mesurer la précarité énergétique, l'ONPE s'appuie sur un panier d'indicateurs : le taux d'effort énergétique, l'indicateur bas revenus et les dépenses élevées, mais aussi le ressenti de l'inconfort, qui est pris en compte comme indicateur du froid et permet de mesurer le phénomène d'autorestriction de la consommation d'énergie.

Les impayés d'énergie, en constante augmentation, ne sont que la partie émergée de l'iceberg : les diagnostics effectués au domicile des ménages en difficulté révèlent bien souvent que les ménages pauvres se privent pour ne pas avoir à régler de trop grosses factures.

auteurs de ce texte sont plus que louables, les difficultés soulevées par les mesures proposées et les doutes qui peuvent naître quant à leur efficacité me font penser que, plutôt que d'inventer des dispositifs nouveaux qui s'avèrent complexes, juridiquement hasardeux et techniquement impossibles, nous serions mieux inspirés de chercher à améliorer les dispositifs existants.

D'abord, il faut se concentrer sur l'état des logements : leur performance thermique est généralement mauvaise, voire exécrable. Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, souvent vétustes, contribuent également à gonfler la facture énergétique des plus pauvres, surtout dans le parc privé. Pour lutter contre la précarité énergétique, un premier enjeu est d'aider les ménages modestes à réduire leur consommation grâce à la réalisation d'opérations d'économies d'énergie dans leur logement. Le Gouvernement- Mme la secrétaire d'État l'a rappelé -a tout à fait conscience de l'urgence que revêt l'accélération de la rénovation énergétique des logements. Le plan de rénovation énergétique des bâtiments, lancé en 2018 par le ministère chargé du logement et le ministère de la transition écologique et solidaire, doit permettre, avec l'appui des financements apportés par le Grand Plan d'investissement, d'augmenter les aides à la rénovation énergétique des logements pour les ménages modestes et très modestes : 1,2 milliard d'euros ont été réservés à cet effet jusqu'en 2022. De nombreux dispositifs ont été mis en place pour accompagner les ménages modestes dans le financement des travaux d'isolation thermique et de rénovation des systèmes de chauffage.

la TVA à taux réduit pour les travaux et les programmes complémentaires financés par les collectivités locales. Afin de faciliter l'accès des ménages modestes qui sont propriétaires occupants de leurs logements à ces financements, qui se multiplient, le Gouvernement a souhaité que les aides versées dans le cadre du CITE et du programme « Habiter mieux » soient fusionnées dans une prime unique dès le 1 janvier 2020. Par ailleurs, à l'occasion de sa prorogation, l'éco-PTZ a été rendu plus opérationnel et fortement simplifié, dès mars 2019 : la condition du bouquet de travaux qui permet de lever la contrainte de liquidité pesant sur les ménages qui ne réalisent pas de bouquet de travaux. Les locataires doivent également pouvoir bénéficier de logements performants. À ce titre, le CITE sera étendu aux propriétaires bailleurs. L'ANAH continuera à soutenir financièrement les propriétaires bailleurs s'engageant à louer leurs logements aux ménages modestes selon les tarifs conventionnés. De même, il convient de saluer l'ambition du Gouvernement de faire de la lutte contre les passoires thermiques une réalité, notamment pour les logements occupés par des ménages aux revenus modestes. À cet égard, l'ambition portée par le plan de renouveau du bassin minier est exemplaire, avec un objectif affiché de rénovation de 23 000 logements dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

la rénovation thermique des logements. Je voudrais également mettre l'accent sur le chèque énergie, qui permet aux ménages bénéficiaires de régler leur facture d'énergie, quel que soit leur moyen de chauffage. Ceux-ci peuvent également l'utiliser pour financer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Le chèque énergie a remplacé en 2018 les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Il permet de pallier les défauts constatés des tarifs sociaux, dont le nombre de bénéficiaires était nettement inférieur à celui des ayants droit. Pour rappel, la valeur moyenne du chèque énergie est passée de 150 euros en 2018 à 200 euros en 2019. Son public a également été élargi, puisque le nombre de ménages concernés est passé de 3,6 millions à 5,8 millions. Nous pouvons imaginer que ce dispositif continuera d'augmenter dans son montant, mais aussi par le nombre de ménages concernés

quant à leur financement possible et, par conséquent, à leur capacité à investir et à procéder à la rénovation thermique nécessaire. Il faudra également mobiliser l'ensemble des propriétaires privés de notre pays pour effectuer

la proposition de loi de notre collègue Fabien Gay nous permet de débattre d'un sujet qui représente, bien entendu, un enjeu social, mais n'en est pas moins un sujet économique et environnemental qui touche au quotidien de nombreux Français.

de 4,5 %. Selon ces critères, un ménage sur cinq est en situation de vulnérabilité énergétique. Par ailleurs, on remarque que les habitants des zones rurales, en particulier les retraités modestes, sont surreprésentés dans ces résultats. En effet, sur 3,8 millions de ménages en situation de précarité énergétique en France, plus de 50 % habitent en zone rurale ou dans une agglomération de moins de 20 000 habitants. En outre, les factures de chauffage dans les zones rurales seraient supérieures de 23 % à la moyenne nationale. Ainsi, il apparaît nécessaire d'accorder une attention particulière à la précarité énergétique en zone rurale. Ce sujet fondamental nous oblige à être pragmatiques et concrets. Tout d'abord, les données que j'ai évoquées justifient la nécessité d'encourager les travaux de rénovation énergétique dans les territoires

des dispositifs existants plutôt qu'une consécration de l'énergie au rang de droit fondamental, dispositif sans effet sur la vie quotidienne des Français. Ensuite, il convient d'éviter toute mesure qui irait dans le sens d'une gratuité totale, ou quasi totale, de l'énergie. En effet, cela reviendrait à déresponsabiliser les ménages. Plus globalement, cela semble contraire aux objectifs d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique. Les citoyens doivent rester conscients de leur consommation énergétique. Aussi, les incitations financières nécessitent d'être davantage dirigées vers les économies d'énergie, les changements de comportements et la lutte contre les passoires énergétiques. De plus, plusieurs dispositifs limitant les effets de la précarité énergétique existent déjà. Il semble important d'en mesurer l'efficacité et de leur apporter les améliorations nécessaires. À ce titre, les tarifs sociaux de l'énergie ont été remplacés en 2018 par le chèque énergie, d'un montant moyen de 150 euros, dont 3,6 millions de ménages ont été destinataires. En 2019, le montant moyen de ce chèque a été porté à 200 euros en moyenne et étendu à 2,2 millions de nouveaux bénéficiaires. Néanmoins, 900 000 personnes ne savent toujours pas qu'elles sont éligibles à ce dispositif et seuls 75 % de ses bénéficiaires profitent profitent réellement de cette aide. Ce dispositif doit être plus visible et sans doute être revalorisé. Plusieurs dispositifs légaux protègent les ménages modestes. Je pense notamment à la trêve hivernale des coupures d'énergie et aux organismes qui aident au paiement des factures d'énergie, comme le fonds de solidarité pour le logement, ou encore les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. La meilleure façon d'éradiquer la précarité énergétique n'en reste pas moins la rénovation des passoires énergétiques. En effet, 80 % des Français seraient logés dans des bâtiments très énergivores. Une forte mobilisation des pouvoirs publics est donc indispensable pour remédier concrètement à ce problème. D'autres dispositifs méritent d'être connus et, au besoin, renforcés. Je pense au programme « Habiter mieux » de l'ANAH, qui permet de subventionner jusqu'à 50 % des travaux pour les ménages modestes. Les certificats d'économies d'énergie pourraient également constituer une piste d'action à renforcer et à élargir. Nous serons également très attentifs aux résultats du plan de rénovation énergétique des bâtiments lancé en 2018 ; il est important de le dynamiser et de l'amplifier pour atteindre les objectifs fixés. La précarité énergétique est donc bien un problème global aux multiples facettes ; sa résolution passera inéluctablement par la simplification, le renforcement et la lisibilité accrue des aides et des processus de rénovation énergétique. Le groupe Les Indépendants ne votera donc pas en faveur de cette proposition de loi, qui ne s'inscrit pas suffisamment dans l'amélioration et le renforcement des dispositifs existants, même si les intentions de ses auteurs sont louables

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la fracture sociale et la précarité sont une réalité dans notre pays. Certains de nos concitoyens souffrent de pauvreté énergétique : on estime qu'environ 12 millions d'entre eux sont touchés Selon des études publiées en mai 2017 par divers instituts, cette situation doublerait le risque d'être en mauvaise santé. La précarité énergétique désigne la difficulté à se chauffer correctement et à un coût acceptable. Elle est causée par des revenus trop faibles pour payer des factures qui augmentent régulièrement. La mauvaise performance énergétique des logements aggrave la situation de personnes en condition de fragilité sociale. Les foyers modestes peinent à payer les factures et doivent renoncer à un certain confort. Le sentiment d'avoir froid chez soi, de se sentir mal chauffé, est un indicateur de précarité énergétique. Celle-ci impacte la facture d'énergie, mais aussi la qualité de vie des personnes qui la subissent. Elle touche des publics divers- des jeunes, des retraités, des familles monoparentales et certains autres foyers - ; on peut donc être touché à tout âge et dans des situations variées. Les chiffres sont éloquents : 87 % des foyers en situation de précarité énergétique sont dans le parc privé ; 70

disent avoir du mal à payer leur facture d'électricité ; les locataires sont trois fois plus concernés que les propriétaires. Enfin, selon une étude de l'Ademe, les 5,5 millions de ménages français les plus modestes consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques, contre seulement 6 % pour les plus aisés. La mauvaise qualité thermique du parc de logement français induit la précarité énergétique : les trois quarts du parc de logement se situent dans les classes D, E, F ou G. Les augmentations de prix aggravent cette situation. Ce problème écologique a aussi un impact social : les propriétaires qui ont les moyens d'acquérir un logement un bâtiment à basse consommation, dit « BBC », logement en moyenne 15 % plus cher qu'un logement traditionnel, ne sont pas touchés par la précarité énergétique, car leur domicile est moins énergivore qu'un logement standard. un tel logement à énergie passive ou positive est quasi introuvable à la location. Certaines solutions innovantes devraient devraient permettre d'éradiquer le fléau qu'est la précarité énergétique. Les bâtiments vieillissent toujours plus et ne peuvent garantir une efficacité énergétique optimale. Rénover le parc des bâtiments permettrait d'endiguer ce problème : il s'agit de faire des travaux de rénovation sur l'ensemble du parc résidentiel, qu'il relève de particuliers, de bailleurs sociaux ou de syndicats de copropriétés. La solution est de mettre en place et de financer un grand plan de rénovation énergétique des logements. Ces rénovations doivent être ambitieuses et ne pas concerner uniquement le remplacement des fenêtres ou le changement des chaudières. Une autre piste concerne les logements mis en location. Pour en finir avec les passoires énergétiques, il faudrait mettre en place une réglementation plus contraignante pour les bailleurs : les logements qui ne respectent pas un standard minimal de performance énergétique devraient être considérés comme impropres Cependant, il est important d'associer à un tel plan des outils de financement incitatifs et orientés vers les ménages aux revenus modestes. Aujourd'hui, la situation est préoccupante, mais elle pourrait encore se dégrader. En effet, la nouvelle directive européenne sur les règles communes pour le marché de l'électricité, adoptée en juin 2019, pourrait apporter des modifications importantes. ce texte prévoit que les États membres pourront décider d'autoriser les fournisseurs à faire payer des frais de résiliation à leurs clients qui mettront fin à un contrat à prix fixe pour une durée déterminée avant le terme Cela signifierait la fin de la gratuité du changement de fournisseur pour les États qui donneraient de telles autorisations aux fournisseurs d'énergie. Il serait souhaitable que la France protège les consommateurs et conserve le principe de la gratuité du changement de fournisseur. Un autre point qui suscite l'attention des consommateurs français est celui de la hausse du nombre des démarchages par les fournisseurs d'électricité. Cela entraîne une augmentation du nombre de litiges portant sur des contestations de souscription ou des dénonciations de pratiques commerciales abusives. Pour les commerciaux employés par les fournisseurs d'énergie, tous les moyens sont bons pour entrer au domicile des particuliers et avoir accès à leurs factures d'énergie. Les méthodes commerciales douteuses sont légion : certains usurpent l'identité de concurrents, ou se font passer pour des releveurs de compteurs. Les personnes âgées sont un public très vulnérable, mais les petites entreprises sont aussi la cible des fausses promesses des démarcheurs. Sans le vouloir,

être à l'origine de la souscription auprès de ce nouveau fournisseur. Pour éviter les dérives de ces démarchages, les fournisseurs d'énergie doivent prendre leurs responsabilités et prévoir un mode de rémunération décent pour les démarcheurs à domicile, avec un salaire fixe complété par une prime variable. Pour garantir le bon fonctionnement du marché de l'énergie libéralisée, plusieurs conditions sont requises : entre autres, les prix des offres de marché doivent demeurer raisonnables et les pratiques des fournisseurs d'énergie doivent être saines. À l'instar de la rapporteure de cette proposition de loi, notre collègue Denise Saint-Pé, que je félicite pour son excellent travail,

à réaliser. De plus, je ne crois pas que le « tout gratuit » soit la bonne solution. Il déresponsabilise et serait trop onéreux pour la collectivité, mais aussi difficile, voire impossible à mettre en oeuvre pour les fournisseurs. Comme l'a préconisé notre rapporteure, il faut améliorer les dispositifs existants, tels que le chèque énergie, avec pour principale cible les plus précaires. C'est pour ces raisons que les membres de mon groupe ne voteront pas cette proposition de loi.

Ces personnes consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d'énergie dans le logement. C'est un problème social qui se traduit par une pauvreté et une solitude croissante de la population. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre pour 2020 explique que la « monorésidentialité » est l'une des causes principales du mal-logement. Cet enjeu social est doublé d'un problème de santé publique et triplé d'un problème environnemental, en raison de la déperdition d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre En effet, si les augmentations des prix de l'électricité et du gaz peuvent impacter les consommateurs et accroître les difficultés qu'ils rencontrent pour payer leurs factures, c'est parce qu'ils occupent des passoires thermiques, des Les pouvoirs publics ont compris l'importance de ce sujet, mais peinent à rénover ces 7 millions de passoires énergivores. La précarité énergétique est donc bien un enjeu fondamental de la transition énergétique.

La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui met ainsi sur la table ce sujet essentiel et vise à compléter les nombreux outils existants au travers de quatre mesures énoncées précédemment. Plusieurs remarques me viennent à l'esprit.

Il me semble donc fondamental de commencer par dresser un bilan des dispositifs déjà existants et de contribuer à leur amélioration. Ensuite, les mesures d'urgence proposées dans ce texte sont curatives et non préventives. Elles risqueraient donc de déresponsabiliser les ménages concernés. En effet, aucune proposition n'est formulée sur le montant de la facture énergétique ou sur les actions à mettre en oeuvre pour maîtriser les consommations et, par conséquent, limiter l'accumulation d'une dette substantielle. de procéder à des coupures d'énergie ne pourrait s'entendre que si des mesures tendant à la maîtrise des consommations et à la rénovation énergétique étaient engagées. Je formulerai la même remarque sur les dispositions fiscales envisagées. la priorité est d'accompagner les ménages précaires de manière préventive, en leur apprenant les bons gestes de consommation et en les mettant en relation avec les services sociaux ou associatifs pour engager des actions de rénovation, par exemple. La réponse durable structurelle à la précarité énergétique, c'est la rénovation du parc immobilier existant, ce qui permettra, au passage, de lutter contre l'artificialisation des sols et de préserver la biodiversité, sujet qui vous est cher, madame la secrétaire d'État, Des investissements accrus permettraient de dépasser les limites des aides actuelles, en finançant mieux des rénovations complètes : chauffage, isolation, ventilation ... Je souligne le rôle déterminant des collectivités locales pour identifier les zones de précarité énergétique et accompagner les ménages. Enedis constitue un vrai soutien. Dans mon département, il a lancé un groupe de travail sur la précarité énergétique avec plusieurs acteurs- collectivités locales, entreprises de proximité et de médiation -et a notamment développé un outil, PrécariTER, qui aide les collectivités à diagnostiquer la précarité énergétique. Avec la question de la simplification des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments, c'est dans la lutte

Les territoires ruraux sont en effet très souvent exposés à ces difficultés, du fait de l'ancienneté des logements et de la sociologie de leur population constituée par un grand nombre de personnes aux faibles revenus- retraités, agriculteurs, contrats précaires, minimas sociaux. Leur mode de chauffage est également plus coûteux : fioul ou électricité. Pour autant, ils en ont assez d'être désignés comme des « délinquants écologiques » au motif que leur empreinte carbone est supérieure à celle d'autres foyers plus aisés, généralement établis en zone urbaine dans un habitat moins énergivore,

Vous le savez, cette situation provoque détresse et colère. Il ne vous a pas échappé, madame la secrétaire d'État, qu'elle a conduit, parmi d'autres raisons, à la crise des « gilets jaunes ». Ceux qui, comme moi, ont, durant plusieurs semaines, eu des échanges avec les manifestants savent combien la revendication d'un meilleur accès à l'énergie ou d'une baisse de ses coûts est prégnante pour certains ménages fragiles. En tant que vice-président de la commission des affaires étrangères, j'insiste aussi sur le fait que la situation pourrait encore s'aggraver si les tensions géopolitiques perduraient, qu'il s'agisse de la crise avec l'Iran et de ses conséquences dans tout le Golfe, des tensions avec la Russie, exportatrice d'hydrocarbures, ou encore de l'escalade militaire en Méditerranée orientale, justement à propos de de l'accès à des ressources énergétiques. Situation sociale nationale dégradée, contexte international explosif : tout concourt à un certain pessimisme. J'ajoute que les difficultés actuelles de la filière nucléaire française ne sont pas une bonne nouvelle pour le consommateur.

et très largement aux dépens des foyers les plus modestes. Cela se confirme de nouveau sur cette problématique énergétique. Madame la secrétaire d'État, mettez les moyens nécessaires budgétaires et fiscaux au service de cette cause.

Cette fiscalité appliquée au taux de 20 % sur la consommation d'énergie est donc particulièrement pénalisante pour les populations les plus fragiles et figure au rang des principales causes qui peuvent faire basculer des ménages dans la précarité énergétique. Les dépenses d'énergie étant des dépenses contraintes, c'est la double peine pour ces ménages dont les factures d'énergie représentent, depuis plusieurs années, une part toujours croissante du budget. Cette fiscalité régressive appliquée à la consommation d'énergie est donc punitive pour ceux de nos concitoyens dont les revenus sont faibles. Elle l'est d'autant plus qu'elle s'applique également aux taxes. Cette double taxation- une taxe sur une autre taxe -représente des enjeux financiers considérables, comme le souligne à juste titre l'UFC-Que Choisir Les particuliers ont payé l'année dernière, rien que sur l'énergie, 4,6 milliards d'euros de TVA sur les taxes. Sur chaque litre d'essence, ce sont ainsi 14 centimes d'euros qui sont payés en TVA sur la TICPE.

que la réduction du taux de TVA est particulièrement utile pour les ménages en situation de précarité énergétique. Pour cette raison, nous proposons de limiter la réduction du taux de TVA sur une première tranche de consommation, dite « de première nécessité », aux seuls aux seuls bénéficiaires du chèque énergie, c'est-à-dire à ceux qui sont le plus en difficulté.

La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur cet amendement pour trois raisons. Premièrement, cette solution reviendrait à faire de la redistribution avec un outil inadapté, celui de la fiscalité indirecte, là où des aides directes ciblées sur les ménages les plus en difficulté seraient bien plus efficaces et bien plus simples à mettre en oeuvre. mesure serait contraire au droit européen, qui permet bien d'appliquer des exonérations totales ou partielles ou des taux réduits aux consommations énergétiques de tous les ménages, mais non d'appliquer des taux différents selon les revenus des consommateurs. Troisièmement, en plus d'être contraire au droit européen, cette mesure présente un fort risque de non-conformité à la Constitution. En effet, il est prévu de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la tranche de consommation qui bénéficierait du taux de TVA réduit. Or l'article 34 de la Constitution précise que c'est la loi qui doit « fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Si cet amendement était adopté, ce serait le pouvoir réglementaire qui fixerait l'assiette et non plus le législateur. Pour alléger la facture énergétique des ménages, je suis convaincue qu'il vaudrait mieux travailler à l'amélioration des dispositifs existants, qu'il s'agisse de soutenir la rénovation énergétique des logements ou d'aider au paiement des factures. Parmi ces aides, je pense en priorité au

des « gilets jaunes ». Cette fiscalité régressive est particulièrement punitive pour les ménages les plus fragiles, qui subissent une double peine. Si, pour Mme le rapporteur, il faut mobiliser d'autres outils redistributifs pour corriger les effets négatifs de ce type de fiscalité,

ne compensera même pas entièrement les dernières hausses des prix de l'électricité, n'infirmera pas ce constat. Force est donc de souligner que ce sont les plus pauvres qui contribuent proportionnellement le plus. Ce n'est pas tolérable. Je rappelle également que, pour protéger l'industrie et éviter le phénomène de fuites de carbone, la loi de finances prévoit d'exonérer les entreprises électro-intensives de certaines taxes.

La surtaxation est aujourd'hui inacceptable et elle n'est plus acceptée. Vous organisez, sous l'autorité du Président de la République, une Convention citoyenne sur le climat, avec un tirage au sort de 150 participants.

Nous sommes là face à une situation d'urgence énergétique et sociale. La lutte contre la précarité énergétique doit être au coeur des politiques de lutte contre la pauvreté et

Cela pourrait à la rigueur se comprendre, si, dans le même temps, ils apportaient d'autres solutions, défendaient d'autres amendements, avançaient d'autres propositions, afin de mettre en accord leurs actes et leur discours. ils sont des millions de Français à souffrir du froid. Ils sont des millions à vivre dans des passoires énergétiques. Ils sont des milliers à avoir des difficultés à payer l'énergie. Ils sont des milliers à devoir choisir entre se chauffer ou se nourrir. Double peine, dit-on. Triple peine ?

les moins responsables du changement climatique. Ce n'est pourtant pas faute d'entendre les alertes lancées par la Fondation Abbé Pierre, l'Observatoire des inégalités ou l'Insee, qui constataient encore récemment que

Je regrette sincèrement qu'aucune suite ne lui soit donnée par la majorité sénatoriale, en réponse à cette véritable urgence sociale qu'est la précarité énergétique. La

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 10 avril dernier, 248 parlementaires de tous bords ont signé la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris,

d'abord par les caractéristiques d'ADP. Ce groupe détient 13 aéroports franciliens et des participations dans 26 aéroports de 30 pays différents.

ADP rapporte 342 millions de dividendes par an, dont la moitié pour l'État, et est propriétaire de 6 680 hectares d'infrastructures et de terrains et de 355 hectares de réserves foncières dédiées à de futures activités immobilières. ensuite par le fait qu'ADP représente un enjeu de portée nationale en matière économique, sociale, stratégique, en termes de mobilités, d'aménagement du territoire et de protection des populations et de l'environnement. Grâce à cette initiative, pour la première fois, la procédure du référendum d'initiative partagée a été engagée pour permettre, en ces temps d'exigences démocratiques toujours plus fortes dans notre société, à nos concitoyens de décider, avec l'intelligence qui les caractérise, du devenir des biens et des richesses de la Nation. Au-delà du débat sur le bien-fondé ou non de cette privatisation, il s'agissait- et il s'agit toujours, et avant toute chose -de laisser enfin aux citoyens la possibilité de décider de l'avenir d'une infrastructure essentielle.

Monsieur le secrétaire d'État, devons-nous, dès à présent, prévoir la mise en place d'une telle instance sur la privatisation d'ADP d'ici à deux ou trois ans ? De nombreux travaux et contre-exemples étrangers, mais surtout le sentiment d'abandon d'une partie toujours plus importante de nos concitoyens, nous invitent à réfléchir à la réduction comme peau de chagrin de notre secteur public, au désengagement de l'État de toutes ses activités stratégiques au profit d'actionnaires privés, dont le seul horizon est la rentabilité à court terme. nous invitent à agir contre l'abandon de toute volonté de s'appuyer sur un secteur public fort pour développer une politique économique et sociale au service du plus grand nombre, sur tout

des privatisations de cette ampleur ne peuvent être décidées par des technocrates nourris aux dogmes de la concurrence libre et non faussée, au nom de la compétitivité, de retours financiers à court terme, du versement toujours plus important de dividendes à des actionnaires avides et peu enclins

Certes, cette procédure référendaire exige un nombre de signatures démesuré puisqu'il doit correspondre à 10 % des électeurs, soit 4 717 396 signatures.

sur l'exercice de ce droit constitutionnel soit fournie à l'ensemble de nos concitoyens, et ce malgré de nombreuses sollicitations. Je dis « droit constitutionnel », car cette procédure référendaire est encadrée par l'article 11 de la Constitution. La validation par le Conseil constitutionnel de la proposition de loi référendaire originelle, déposée par 248 parlementaires, ouvre un droit constitutionnel : celui d'apporter son soutien à la tenue d'un référendum. En ce sens, ce droit s'apparente au droit de vote. Il ne s'agit en rien d'une simple pétition, contrairement à ce qu'affirment souvent le Gouvernement et ses soutiens. Je le répète : il s'agit de mettre en oeuvre l'article 11 de la Constitution. En démocratie, les citoyens doivent être informés de la possibilité d'exercer un tel droit. L'État doit affecter des moyens en ce sens,

doit ainsi intervenir auprès des chaînes publiques d'information, qui ont un rôle citoyen à jouer en la matière, afin qu'elles diffusent largement l'information sur ce sujet. C'est cela le respect du pluralisme, fondement de tout État démocratique

Radio France a refusé de diffuser les communiqués financés par les parlementaires eux-mêmes, sur leurs deniers personnels. Que dire encore des mairies qui n'ont pas mis en place de bureau d'aide pour que les citoyens puissent apporter leur soutien au RIP alors qu'elles y sont obligées par la loi, sans être aucunement inquiétées ? inquiétées ? C'est la loi, monsieur ! Que dire enfin du refus de la Commission nationale du débat public (CNDP), dont c'est pourtant la vocation, d'organiser un débat sur le projet de privatisation d'Aéroports de Paris, en complément du projet de référendum d'initiative partagée ?

malgré les dysfonctionnements du site internet, malgré le silence assourdissant des grands médias et du Gouvernement, malgré l'absence de campagne officielle, plus d'un million de personnes ont apposé leur signature pour la tenue

un soutien fort aux services publics- hôpitaux, écoles ou transports. Ils exigent des droits démocratiques réels sur les questions concernant la société tout entière et un contrôle sur les biens communs et les services publics. Mais plus que la question de la maîtrise des biens communs, ce sont les limites de la monarchie républicaine qu'est le régime présidentialiste de la V République et la méfiance croissante des citoyens envers la démocratie représentative, qui sont aujourd'hui en jeu. Le RIP est une occasion constitutionnelle historique de redonner du souffle à notre démocratie en améliorant cette procédure de démocratie participative. Alors que se déroule dans notre pays un mouvement social sans précédent, Emmanuel Macron a tort de ne pas écouter le peuple de France, sur cette question comme sur d'autres. À aucun moment, sauf lorsqu'il câline sa majorité parlementaire, il ne lui envoie de signaux apaisants et rassembleurs. Il préfère s'enfermer dans une posture qui illustre bien les dérives d'un pouvoir à bout de souffle, pétri de certitudes, dans un système institutionnel vermoulu,

une opposition bête et méchante, un accro à la légitimité de la chose votée, peut-être même une atteinte aux prérogatives du Parlement, en tout cas un crime de lèse-majesté

qu'il méprise les corps intermédiaires, voire le Parlement. Avec cette démarche, nous l'avons pris au mot. « Qu'ils viennent me chercher ! », avait-il dit. Nous sommes là ! Et beaucoup de Français sont à nos côtés.

d'abord, parce qu'on va brader un bien de l'État qui rapporterait plus en le gardant pendant les soixante-dix ans de l'éventuelle prochaine concession ; économique ensuite, parce que Roissy et Orly sont les portes d'entrée de la France en termes de tourisme, et il est important que la puissance publique garde la main ; environnementale enfin, parce que l'aménagement et le développement aérien sont des questions qui préoccupent préoccupent pour l'avenir- là encore, l'État doit pouvoir intervenir pour réguler. La décision de privatiser a un impact national qui légitime un référendum sur tout le territoire. Je le concède, monsieur le secrétaire d'État, ce n'est pas le seul sujet de préoccupation des Français. Il y en a bien d'autres qui ruissellent en ce moment : assurance chômage, pouvoir d'achat, retraites ... Ils sont divers. Mais ils ont un point commun : la morgue avec laquelle le Président de la République, vous-même et votre gouvernement accueillez les craintes de nos concitoyens. Refuser ce référendum serait porter un coup de plus à notre démocratie. Nous vous proposons une soupape, un moyen d'échanger avec le pays. Opposer une fin de non-recevoir à cette demande n'est pas une méthode. Ce serait de la provocation ; une de plus, me direz-vous À les multiplier, vous faites le lit du populisme et vous portez atteinte à ce qu'il y a de plus sacré dans notre République : l'exigence démocratique, qui repose sur la souveraineté du peuple

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la privatisation d'Aéroports de Paris est assurément un des grands points d'achoppement de ce quinquennat. Annoncé en 2018 et inscrit dans la loi Pacte, adoptée l'an dernier, le processus est depuis lors mis entre parenthèses par le déclenchement, pour la première fois, de la procédure référendaire dite « d'initiative partagée », après le dépôt au mois d'avril 2019 d'une proposition de loi signée par plus d'un cinquième des parlementaires, dont votre serviteur. Les privatisations ou ouvertures de capital d'entreprises publiques en France ne datent pas d'hier. Commencées en 1986 sous la première cohabitation, elles ont été poursuivies depuis par presque tous les gouvernements, sauf pendant la crise financière des années 2008-2009, où la chute des valeurs boursières les avait rendues peu rentables. Parmi des privatisations restées emblématiques, on peut rappeler celles de TF1, de grandes banques, de Total et d'Usinor-Sacilor dans les années 1980 et au début des années 1990, l'ouverture du capital de Renault en 1996 et de France Télécom à partir de 1997, déjà de certaines compagnies d'autoroutes, d'EDF-GDF à partir de 2005 et, plus récemment, la baisse des participations de l'État au capital du groupe Safran. L'ouverture du capital d'ADP a, quant à elle, débuté sous le gouvernement Villepin. Dans les années 2010, ce sont les grands aéroports régionaux qui ont connu à leur tour une vague de privatisations : l'aéroport de Toulouse, dans les conditions que l'on sait, et ceux de Lyon et de Nice. ADP n'est pas une société anodine. Créée à la Libération, elle a accompagné la formidable modernisation de l'économie française pendant les Trente Glorieuses, avec l'ouverture d'Orly en 1961, puis de Roissy en 1974. C'est aujourd'hui le premier groupe de gestion aéroportuaire au monde en nombre de passagers, avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et un résultat net positif de 600 millions d'euros en 2018. Sa filiale à l'international gère 24 aéroports répartis dans 13 pays différents, dont l'Algérie et la Turquie. Le chapitre de la loi Pacte consacré aux privatisations semble faire peu de cas de cette histoire et de cette situation exceptionnelle, en traitant pêle-mêle de sujets aussi divers qu'ADP, la Française des jeux ou Engie. Sans mépris aucun pour ces dernières entreprises, on doit pourtant bien reconnaître que les enjeux d'ADP dépassent très largement ceux des jeux de loterie ou de la prévention. Il s'agit pour l'État français d'une question stratégique et patrimoniale. D'une certaine manière, ce qui se joue ici, c'est l'identité économique de la France. Le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de nos textes fondamentaux au même titre que la Déclaration des droits de l'homme dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est bien le cas d'Aéroports de Paris, qui joue de plus le rôle stratégique de principale porte d'entrée sur le territoire national. L'an dernier, lors de l'examen de la loi Pacte, le Sénat avait majoritairement rejeté les articles de privatisation, à l'occasion d'une rare alliance entre la droite et la gauche de cet hémicycle. Le groupe du RDSE avait très majoritairement approuvé ces suppressions. Aujourd'hui, les Français restent aussi majoritairement opposés à une telle mesure. Comment dès lors expliquer les difficultés pour réunir le nombre nécessaire de signatures pour soumettre à référendum l'objet de la proposition de loi ? À l'évidence, les conditions prévues par l'article 11 de la Constitution apparaissent trop restrictives : un dixième du corps électoral, soit 4,7 millions de citoyens, cela équivaut à un score d'environ 20 % aux dernières élections, score que certaines formations ont d'ailleurs eu du mal à atteindre. À titre de comparaison, les pays qui ont réellement mis en pratique ce mode de consultation ont retenu des seuils bien plus bas. L'exemple suisse est bien connu les référendums à l'échelle fédérale nécessitent la signature de 100 000 citoyens, soit moins de 3 % du corps électoral. En Italie, le seuil est fixé à 500 000 électeurs, bien au-dessous des 4,7 millions nécessaires chez nous, pour une population équivalente. Beaucoup d'interrogations demeurent à propos de ce dossier. Par exemple, la difficulté à trouver des informations précises sur le Fonds pour l'industrie et l'innovation, que ces cessions de participations sont censées financer. Par ailleurs, si je ne nie pas l'intérêt des projets annoncés, ceux-ci masquent encore mal l'absence d'une réelle politique industrielle en France et en Europe. Enfin, le risque de le risque de hausse des redevances aéroportuaires, comme dans le cas des concessions d'autoroutes, et les conditions d'indemnisation des futurs actionnaires dans l'éventualité d'une fin de concession anticipée continuent de susciter de réelles interrogations, en particulier sur les conséquences sur le budget de l'État et pour d'autres acteurs, comme les compagnies aériennes, ainsi que sur le risque de suppression des petites lignes Paris-province non rentables. C'est pourquoi, pour répondre à la question peut-être un peu rhétorique de mes collègues du groupe CRCE, l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris continue à mes yeux d'être une exigence démocratique. La parole

privatiser ADP, c'est repenser la place de l'État au XXI siècle : il s'agit de passer d'un État rentier à un État investisseur, un État stratège qui investit pour l'avenir des Français. Le produit des cessions doit abonder un fonds d'innovations de rupture doté de 10 milliards d'euros, nécessaire à notre économie nationale : stockage de l'énergie, intelligence artificielle, robotique L'État stratège n'est pas nécessairement un État actionnaire de toutes les entreprises. Le fonds d'innovation doit permettre de préserver la souveraineté du pays, pour que notre économie ne dépende pas uniquement de brevets et de licences de l'étranger. Il faut aussi garder à l'esprit que de nouveaux investissements sont nécessaires, par exemple pour la construction d'un quatrième terminal. C'est parce qu'ADP se porte bien qu'il a de nouveaux besoins de financement ; sa forme actuelle ne lui permet pas de les obtenir. Par ailleurs, un tiers des bénéfices d'exploitation d'ADP provient de l'activité aéroportuaire, mais les deux tiers proviennent des boutiques de luxe, des hôtels et des parkings. Ce n'est pas le rôle de l'État de percevoir des dividendes liés à ces activités Le groupe ADP est international. Il est présent dans plus de trente pays et détient par exemple des participations dans les aéroports d'Amsterdam et d'Istanbul. Il s'agit de conforter une stratégie de consolidation à l'international déjà engagée par le groupe pour s'imposer parmi les leaders mondiaux. ADP perçoit la cession de la participation publique comme une aide dans sa stratégie. La cession des participations publiques a pour objectif l'entrée de nouveaux investisseurs qui permettront d'emmener le groupe aux plus hauts niveaux et de le conforter comme leader mondial. Ce transfert au secteur privé est évidemment assorti de plusieurs garde-fous législatifs pour que l'État conserve ses prérogatives en matière d'autorisation d'investissements. En effet, la reprise du contrôle des actifs par l'État sera opérée au bout de soixante-dix ans. Pendant cette période, les actifs sont incessibles sauf autorisation expresse de l'État. De plus, des enseignements ont été tirés des erreurs commises lors de la conclusion des concessions autoroutières. Des contrats de régulation économique pluriannuels seront renégociés tous les cinq ans entre l'État et ADP. Concernant les salariés, le régime applicable ne sera pas affecté par la privatisation. Cette garantie inscrite dans la loi fait d'ailleurs suite à un amendement communiste adopté à l'Assemblée nationale. Ce dispositif apparaît plus efficace qu'une concession classique, qui aurait imposé une mise en concurrence, puis la conclusion d'un contrat avec l'opérateur retenu et qui n'aurait pas permis à l'État de garder un contrôle aussi important que celui qu'il aura dans le cadre de la privatisation d'ADP. En outre, une concession classique aurait conduit à une hausse des redevances aéroportuaires avec une répercussion sur les compagnies aériennes. Or, dans le cadre du contrat de régulation économique pluriannuel, les compagnies sont associées pour le niveau de redevances. niveau de redevances. La sécurisation de la frontière et la régulation du trafic- cela inclut les horaires de décollage pour les communes aux alentours -restent gérées par l'État. Il est à noter que le Gouvernement a même renforcé la police aux frontières voilà un an. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, la privatisation d'ADP semble nécessaire. Faisons donc un référendum ! Cet avis n'est pas partagé par un certain nombre de nos collègues parlementaires. Ceux-ci ont choisi de déclencher un projet de référendum d'initiative partagée Le référendum d'initiative partagée est le dispositif prévu, depuis la révision constitutionnelle de 2008, à l'article 11 de la Constitution. Celui-ci prévoit qu'un référendum peut être organisé « à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». À ce jour, au moins 185 parlementaires ... 248 ! ... issus de plusieurs partis d'opposition soutiennent ce projet de référendum. Le Conseil constitutionnel a en outre donné son feu vert à ce projet. Cependant, il n'en va pas de même concernant la troisième condition, puisque la pétition en ligne recueille un peu plus d'un million de signatures sur les 4,7 millions que requiert le RIP, ... Vous avez essayé de S'il n'est pas question ici de discuter de l'utilisation du référendum d'initiative partagée, qui est un droit constitutionnel, le déclenchement du projet de RIP pour contester la privatisation d'ADP est, lui, sujet à caution.

nous incarnons ici. Il est cependant à craindre, au-delà du cas particulier d'ADP, que l'initiative de nos collègues puisse ouvrir une brèche susceptible de fragiliser le système de représentation politique. Jusqu'à présent, la mise en oeuvre du RIP, inscrit dans la Constitution en 2008, paraissait suffisamment exigeante pour que la procédure ne soit utilisée que dans des circonstances exceptionnelles.

poursuivre, monsieur Théophile. La France a un besoin évident de renouveau démocratique et d'une plus grande participation directe des Français aux choix politiques, notamment sur le plan local. Le mouvement des « gilets jaunes » en a souligné l'urgence. En définitive,

risque de devenir la plus grosse de l'histoire française, nos concitoyennes et concitoyens ne bénéficient d'aucune information officielle leur permettant de donner leur avis. C'est un déni démocratique, mon cher collègue Théophile ! Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour qu'une campagne d'information soit lancée, ce qui n'a malheureusement pas abouti, en tout cas jusqu'à présent.

Plus de 38 400 personnes se sont exprimées, soit pratiquement 5 % des électeurs. Sur la France entière, ce sont plus d'un million de personnes qui exigent la tenue d'un référendum sur la privatisation, ou non, du groupe du groupe ADP. Je tiens à ce propos à saluer les actions que nous avons menées, comme à la Fête de l'Humanité au mois de septembre dernier sur l'initiative de notre groupe, ou encore lors du meeting organisé au mois de juin dernier à la Bourse du travail de Saint-Denis l'initiative de mon collègue député Stéphane Peu, qui réunissait des parlementaires de toutes sensibilités politiques, du PCF au PS, en passant par la France insoumise, Les Républicains, Génération.s et Europe Écologie Les Verts. Sans compter les dizaines d'actions sur nos territoires. Les enjeux sont majeurs. pense tout d'abord aux conséquences économiques. En moyenne, Aéroports de Paris rapporte 170 millions d'euros de dividendes chaque année à l'État. En cas de privatisation, non seulement cette source de revenus disparaîtrait, mais, en plus, l'État devrait s'acquitter d'indemnisations supplémentaires particulièrement vertigineuses : près d'un milliard d'euros pour indemniser financièrement les actionnaires minoritaires actuels, qui risqueraient, après les soixante-dix ans de privatisation prévus par la loi, d'être expropriés pour une nouvelle nationalisation, alors alors même qu'il est également prévu que l'État rachète son dû dans soixante-dix ans. Ainsi., l'État y perdrait triplement : un milliard d'euros d'indemnités en faveur des actionnaires minoritaires ; 170 000 euros de bénéfices en moins par an, c'est-à-dire presque 12 milliards d'euros sur soixante-dix ans ; et, bien entendu, le prix qu'il faudrait payer pour racheter ADP dans soixante-dix ans ! Monsieur le secrétaire d'État, quand on cherche de l'argent : là, il y en a ! C'est à l'encontre de tout bon sens, alors même qu'ADP est une entreprise rentable qui offre de nombreuses perspectives prospères pour l'avenir, comme le laissent présumer le nouveau terminal 4 à Roissy, prévu pour 2025, ou les récents aménagements de l'aéroport d'Orly. Le Gouvernement prétend vouloir investir dans un fonds pour l'innovation grâce aux recettes de cette privatisation. Les recettes annuelles d'ADP, en constante hausse, ne pourraient-elles financer ce fonds sur plusieurs années ? Le deuxième enjeu capital soulevé par la privatisation d'ADP est politique. Comme le rappelle le professeur de droit public Paul Cassia, cette opération soulève un problème relevant de la souveraineté même de l'État français. En effet, plus de 100 millions de passagers transitent chaque année par cette plateforme pour entrer sur le territoire ou en sortir, faisant d'ADP la plus grande frontière française. Pas moins de 80 % des visiteurs étrangers passent par ADP, qui possède donc des infrastructures sensibles Privatiser ces infrastructures signifie nécessairement menacer la capacité de l'État à contrôler intégralement et sans intermédiaire les entrées et sorties du territoire, qui vont dépendre dépendre de son dialogue avec un groupe privé. Un troisième enjeu particulièrement important est le risque d'anticonstitutionnalité d'une telle privatisation. En effet, cette opération entre directement en contradiction avec le neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » C'est sur cette base que le législateur avait déjà refusé la privatisation d'ADP en 2005. Cette Cette privatisation potentielle soulève également un enjeu fort lié aux risques de suppressions d'emplois et de précarisation d'une partie des salariés d'ADP. Pour rappel, près de 90 000 salariés travaillent à Roissy et plus de 25 000 à Orly, sans compter les emplois induits. Et que dire de l'enjeu écologique d'une telle privatisation à une époque où nous subissons directement les conséquences du réchauffement climatique ? Que dire des conséquences sur la vie des riverains ? Je pense particulièrement aux nuisances sonores ! Il est à craindre qu'une privatisation d'ADP n'aggrave la situation, en intensifiant le trafic aérien et en remettant en cause le couvre-feu actuel, qui interdit le survol des avions entre vingt-trois du matin. Enfin, une privatisation aboutirait nécessairement à une augmentation des tarifs et à un remaniement qui pourraient menacer certaines lignes, par exemple celles reliant la France hexagonale à ses territoires d'outre-mer. À La Réunion, un collectif d'usagers, Réunion ADP, craint particulièrement les hausses des taxes aéroportuaires, qui correspondent actuellement à 50 % du prix d'un vol. Alors que des milliers d'étudiants ultramarins viennent chaque année faire leurs études en France métropolitaine, comment garantir leur mobilité sans hausse supplémentaire ? Au regard des nombreuses conséquences que je viens d'évoquer, l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris relève d'une exigence démocratique. Il y va du droit des citoyennes et des citoyens à protéger le devenir des biens communs et des services publics. Il y va également du devoir de l'État d'écouter les mobilisations inédites et les nombreuses voix,

Parmi toutes les mesures de bon sens attendues de longue date par les entrepreneurs et les salariés français, une disposition de ce texte cristallisait les tensions politiques. Il s'agissait de la privatisation d'Aéroports de Paris. Un an après, nous nous réunissons de nouveau dans notre hémicycle pour aborder cet épineux sujet. Cependant, l'objectif de ce débat n'est pas de remettre le même ouvrage sur le métier. Car, depuis lors, les termes du débat ont changé. Une proposition de loi référendaire a été déposée contre cette privatisation. La question qui nous est posée aujourd'hui est la suivante : l'organisation de ce référendum est-elle une exigence démocratique ? Nous devons donc définir ce que signifie l'expression « exigence démocratique ». On peut l'entendre de deux façons. D'une part, s'agit-il d'une demande du peuple français suffisamment forte pour justifier l'organisation d'une large consultation ? D'autre part, s'agit-il d'une obligation institutionnelle fondée sur un principe de notre droit par la demande populaire. J'éviterai pour ma part de me poser en porte-voix du peuple français. Je me contenterai de me référer à des critères objectifs. Or nous disposons en la matière d'un baromètre assez précis. En effet, en choisissant la voie du référendum d'initiative partagée, les parlementaires ayant cosigné la proposition de loi référendaire ont sollicité le soutien de nos concitoyens. La proposition ne pourra être adoptée que s'ils parviennent à réunir les signatures de 10 % du corps électoral, soit quelque 4,7 millions de Français, dans les neuf mois suivant le dépôt de la proposition. À quelques semaines de l'échéance, les soutiens ne dépassent guère le million de signatures, soit à peine 2 % du corps électoral. Difficile, dans ce contexte, de parler de demande populaire forte viens à l'obligation institutionnelle. Dans le cas où le seuil des 4,7 millions de signatures ne serait pas atteint, la proposition de loi référendaire resterait lettre morte. Dès lors, aucune loi de la République ne pourrait contraindre le pouvoir exécutif à organiser un référendum. En somme, il apparaît qu'un référendum sur la privatisation d'ADP n'a rien d'une « exigence démocratique ». Nos institutions ne nous y obligent pas, et le peuple ne le demande pas. La deuxième question porte sur la décision du Conseil constitutionnel jugeant recevable cette proposition de loi référendaire. Cette décision a suscité de nombreuses critiques, notamment celles, dans une tribune parue le 14 mai dernier dans, de deux constitutionnalistes de renom, qui considéraient que le Conseil constitutionnel avait commis une double faute, à la fois juridique et démocratique, en jugeant recevable cette proposition de loi. Leur argumentation s'appuie notamment sur le fait que cette procédure ne respecterait pas l'esprit de réforme constitutionnelle de 2008 ayant instauré le référendum d'initiative partagée. En effet, une proposition de loi référendaire ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. L'initiative de nos collègues a donc joué sur le calendrier et, pour ainsi dire, sur les mots, en visant à abroger une disposition votée par les assemblées, mais non promulguée par le pouvoir exécutif. Ces critiques ont été entendues par le Conseil constitutionnel lui-même, dont le président a cru nécessaire de justifier sa décision, fait rarissime, en publiant un communiqué. Petite parenthèse : ce communiqué rappelle préalablement que le Conseil constitutionnel a validé la loi Pacte, y compris les articles prévoyant la privatisation d'ADP, ce que l'on oublie trop souvent. J'ai donc été étonné d'entendre dire à l'instant que ces articles étaient anticonstitutionnels. N'en déplaise à ceux qui ont déclenché la procédure de référendum, cette privatisation a donc force de loi, et il y a tout lieu de penser que cela le restera, tant nous sommes loin aujourd'hui des 4,7 millions de signatures. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que, dans le vocabulaire très particulier et très prudent du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius indique qu'il y a « matière à réflexion sur la manière dont cette procédure »- celle du référendum d'initiative partagée -« a été conçue ». conçue ». En français de tous les jours, cela signifie que le législateur s'est pris les pieds dans le tapis en 2008, et Laurent Fabius suggère donc à mots couverts qu'il faudra y revenir lors d'une prochaine révision constitutionnelle. Quelle est en effet la conséquence importante et fâcheuse du texte constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui rédigé ? C'est la faille dans laquelle se sont engouffrés les parlementaires ayant lancé la procédure de demande de référendum un jour avant la promulgation de la loi. Avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on va désormais pouvoir proposer un référendum sur tous les sujets pendant même l'examen de la loi. Cela revient à opposer démocratie directe et démocratie représentative, alors qu'elles étaient jusqu'à présent complémentaires, à opposer au même moment les deux expressions de la volonté nationale que sont le vote des représentants du peuple et le référendum. Dans ces conditions, cette forme de démocratie participative vise moins à compléter les mécanismes de la démocratie représentative qu'à leur faire échec. C'est un problème grave. Il nécessitera, comme je l'ai déjà souligné, une clarification de l'article 11 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle. Si nous ne le faisons pas, nous aurons laissé, nous, parlementaires, discréditer le travail des assemblées en le soumettant aux impératifs de la démocratie plébiscitaire. Et nous connaissons tous l'écueil principal de cette démocratie plébiscitaire : elle conduit les citoyens à se prononcer pour ou contre un gouvernement plutôt que pour ou contre une mesure, aussi importante soit-elle pour le pays. Bien sûr ! Nous sommes au coeur des débats depuis un an sur les rapports de la démocratie représentative et de la démocratie directe. J'ai exprimé à d'autres occasions les graves inquiétudes que m'inspirent les dérives vers la démocratie directe, démocratie d'émotion quand ce n'est pas démocratie de l'émeute Dans les circonstances que traverse aujourd'hui notre pays, et alors que la vague populiste menace un peu partout les régimes démocratiques, ... On l'attendait ! ... il est plus que jamais essentiel de lui résister.

L'accord du Parlement était donc obtenu, dans le plus strict respect des institutions et des principes démocratiques, mais pas nécessairement dans celui de l'opinion publique. Tandis que l'État s'efforçait de diminuer ses dépenses et de consolider ses recettes, l'opinion publique, alimentée par les mouvements sociaux et politiques, s'interrogeait chaque jour davantage sur l'intérêt de vendre des actifs rentables et de renoncer à des rentrées d'argent récurrentes, appauvrissant l'État. Le mouvement des « gilets jaunes », avec ses revendications de justice sociale et de meilleure redistribution des richesses, a rebondi sur le dossier de la privatisation du groupe ADP, perçue comme une « spoliation » du patrimoine des Français, d'autant que les chiffres du groupe explosaient, ADP devenant le numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire en nombre de passagers et le détenteur du premier aéroport de l'Union européenne, Roissy-Charles-de-Gaulle, à la suite du Brexit. En avril dernier, 185 de nos collègues se sont associés pour lancer une première procédure de référendum

Mais existe-t-il une alternative dans le contexte que nous connaissons ? Le vote du Parlement suffit-il encore à légitimer le choix de privatiser ADP face à une

Tout choix politique s'inscrit dans un contexte, mes chers collègues. C'est, me semble-t-il, l'enchaînement des événements de ces derniers mois et les déclarations maladroites de l'exécutif qui, aujourd'hui, confèrent à la consultation des citoyens par référendum une légitimité en quelque sorte supérieure et complémentaire à celle du vote du Parlement. L'argument qui met en avant les 10 % de soutiens nécessaires à l'organisation d'un référendum n'est plus audible après les propos du Président de la République, qui qualifiait de « signal déjà fort » la mobilisation d'un million de signatures. Le référendum sur la privatisation d'ADP est désormais le talon d'Achille du Gouvernement, avec ce dilemme : faut-il prendre le risque de le perdre ou l'esquiver ? Refuser un référendum, c'est discréditer, une fois de plus, la parole du politique. Dans le contexte et avec les menaces que nous connaissons, ce serait vécu comme un nouvel acte de défiance d'un président qui n'écouterait plus les Français, et craindrait même de leur laisser la parole. Le risquer, c'est en revanche se présenter comme le garant d'une démocratie assumée. Je conclurai par une formule souvent employée par le Président de la République : « N'ayez pas peur

Alors que bien des aspects de ce projet allaient dans le bon sens, selon une regrettable habitude, une disposition introduite dans le texte allait polariser l'attention et polluer le débat du début à la fin ... Je veux parler de la privatisation d'ADP. M'appuyant sur les similitudes avec l'expérience récente et cuisante de la privatisation des concessions d'autoroute, qui aurait dû nous instruire utilement sur ce type de procédure, j'étais alors l'un des premiers, avec Fabien Gay, à dénoncer vigoureusement la privatisation d'Aéroports de Paris pour des raisons simples, essentiellement stratégiques, financières, environnementales et sécuritaires sur lesquelles il n'est plus besoin de revenir, tellement le débat a fait rage. En revanche, je n'ai pas fait partie, le 9 avril 2019, des 248 parlementaires, toutes tendances confondues, à l'initiative du lancement de la procédure de référendum d'initiative partagée. Je ne l'ai pas fait parce que, selon moi, pour répondre précisément à la question posée dans ce débat, l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris n'est absolument pas une exigence démocratique Le référendum d'initiative partagée est une forme particulière du processus législatif français. Il associe le corps électoral à une proposition de loi, via un recueil de soutiens.

Le déclenchement de la procédure appartient aux seuls parlementaires, le soutien des électeurs intervenant dans un second temps. De ce fait, le mécanisme ne peut être qualifié de référendum d'initiative populaire, bien que l'expression ait été largement employée pour le désigner. Pour ma part, je constate que ce mécanisme n'est en fait qu'un « alibi de modernité » doublé d'une « course d'obstacles » dont le est décrit aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution. Le remède est pire que le mal Le seul but est en réalité de créer un effet d'annonce dans les médias sur un élan démocratique du système politique, alors que le mécanisme est conçu pour assurer que le référendum n'aboutisse en aucun cas. La proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui, relative au statut d'Aéroports de Paris, en est un criant exemple. Le délai court du 13 juin 2019 à minuit jusqu'au 12 mars 2020 avant minuit. En décembre 2019, nous avons franchi le cap du million de soutiens enregistrés sur le site internet du ministère de l'intérieur. Courage, mes chers collègues, il ne vous reste plus qu'à en trouver 3 millions et demi en un peu plus d'un mois ! Un jeu d'enfant lorsque l'on s'essaie lorsque l'on s'essaie au parcours du combattant nécessaire pour s'enregistrer sur ce fameux site, lorsqu'il fonctionne ... La démocratie représentative doit avoir la « primauté » et « le développement des instruments de démocratie directe ou participative doit avoir pour corollaire le renforcement du rôle du Parlement ». C'est clairement ce qu'a affirmé le groupe de travail sur la révision constitutionnelle, réuni par Gérard Larcher, président du Sénat, le 20 mars 2019. La démocratie directe ou participative est complémentaire de la démocratie représentative, et il n'y a pas lieu d'opposer l'une à l'autre. Les trois propositions du président du Sénat pour revivifier le droit de pétition devant notre assemblée font preuve de sagesse. Premièrement, un droit de tirage citoyen permettrait à des citoyens, une pétition, de déclencher la création, une fois par session, d'une mission d'information sénatoriale.

Mais prenons garde à ce que le rythme de réformes d'opportunité, mineures et précipitées, ne conduise le « mécano constitutionnel », selon l'expression chère au doyen Vedel, à l'emporter sur la logique de l'équilibre institutionnel ! La parole est

figurait pas dans le programme présidentiel. Il est donc tout à fait légitime que les citoyennes et les citoyens de notre pays puissent s'en emparer, notamment via le référendum d'initiative partagée.

et économiques. C'est une hérésie, un contresens historique majeur ! L'intérêt général commande au contraire d'en garder la maîtrise, et les Français veulent prendre part à ce débat. La parole

Notre système démocratique est certes imparfait, mais il permet aux citoyens de s'exprimer régulièrement à l'occasion des scrutins, qu'ils soient nationaux ou locaux.

Nos électeurs savent très bien nous rappeler à nos obligations quand nous nous en éloignons. En voulant favoriser l'accès au référendum sur des sujets techniques et économiques comme la privatisation d'Aéroports de Paris,

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je suis un fervent défenseur des institutions de notre République et de l'existence du Parlement

le 24 octobre 1973, un décret signé du président Pompidou donnait le nom de Charles de Gaulle à l'aéroport de Roissy,

un principe constitutionnel, ce qui aurait sans doute mérité un débat en tant que tel, et non une discussion au détour d'un article d'un texte aussi hétéroclite que la loi Pacte.

mais je reste convaincu qu'Aéroports de Paris n'est pas qu'une question de capitaux, de rentabilité et de technique. Il s'agit d'un équipement stratégique et, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, d'une ambition dont l'État ne peut être absent. Il doit en être acteur.

Je crains que nous n'ayons pris le risque de sacrifier l'avenir en espérant glaner quelques recettes pour boucler un budget toujours déficitaire. Mais s'agissant Mais s'agissant d'ambitions nationales, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement avec l'ampleur du débat qui a eu lieu autour d'un autre aéroport, celui de Notre-Dame-des-Landes, avec ses 180 décisions de justice.

aura 88 ans quand la concession se terminera ! Je crains que le Gouvernement ne tire une traite sur l'avenir.

Si l'on peut et l'on doit s'interroger sur la pertinence économique de cette privatisation, sur sa cohérence stratégique, on ne peut ignorer la problématique politique et démocratique posée par cette cession. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause l'essence même de notre système de démocratie représentative. Mais certaines décisions s'avèrent des symboles si forts que, même légales, même en respectant formellement les prérogatives et votes du Parlement, elles souffrent d'une légitimité tremblante et incertaine. alors qu'ADP est tout sauf un petit aérodrome de province ou une énième zone commerciale de la grande couronne francilienne, l'État a voulu graver son futur dans une sous-section des 221 articles de la loi Pacte. Sept articles- au milieu des modifications sur les formalités administratives, la formation professionnelle, le jour des soldes, les assurances, etc. -résument en quelques mots des orientations clés pour l'avenir du transport aérien, l'aménagement du territoire, la stratégie économique et financière de notre Nation, et même sa souveraineté. final, est de rembourser comptant seulement 0,5 % de la dette publique ... N'oublions jamais qu'un grand aéroport est aussi une porte d'entrée territoriale, un espace frontalier avant d'être une galerie marchande. Ne fallait-il Ne fallait-il pas au moins un projet de loi spécifique ? Évidemment ! Mais vous avez fait un autre choix. Cette volonté de privatisation d'ADP, enfouie au fond de la jungle touffue d'une loi obscure, est révélatrice, sur le fond comme sur la forme, d'une gouvernance lointaine et technocratique qui attise le volcan de l'incompréhension et le magma de la colère chez de nombreux Français. Quand on vend les bijoux de la famille, ce n'est jamais bon signe, et il ne faut pas s'étonner que la famille demande des comptes Les Français veulent un État stratège, pas un gang de boursicoteurs « gagne-petit » leur expliquant doctement qu'ils n'ont rien compris. Les Français ont du bon sens, ils comptent mieux que les ordinateurs de Bercy et ils ont de la mémoire. Ils se souviennent des pathétiques privatisations du réseau d'autoroutes et de l'aéroport de Toulouse. Il est toujours temps de corriger une erreur, ou au moins de fortifier une décision, de la rendre incontestable. Comment ? En donnant la parole au peuple ! Pourquoi le refuser, alors que le Gouvernement ne cesse de proclamer un souci d'écoute et de proximité qui reste tout virtuel ? En avez-vous donc peur, monsieur le secrétaire d'État ? Certains disent que le référendum est un outil dangereux, pernicieux, que les citoyens ne répondent pas vraiment à la question posée, mais en profitent plutôt pour exprimer un rejet. Il fut un Il fut un temps, pas si lointain, à l'aube de la Ve République, où le Président de la République donnait régulièrement la parole au peuple. Certes, n'est pas de Gaulle qui veut Je fais partie des parlementaires qui se sont associés pour déclencher le processus conduisant à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. À ce jour, plus d'un million de nos compatriotes ont signé cette demande, est insuffisant pour imposer le référendum, mais suffisant pour que le Gouvernement entende le malaise exprimé. Monsieur le secrétaire d'État, si vous êtes sûr du bien-fondé de votre décision, je ne doute pas que vous saurez en convaincre les Français. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote », a écrit Charles de Gaulle. Puisse donc le Gouvernement être audacieux, courageux et pédagogue, monsieur le secrétaire d'État ! Puisse le Gouvernement être gaulliste, ou au moins gaullien ! Un référendum lui en donnerait l'occasion.

Je me réjouis de voir que le débat démocratique est toujours bien vivant, puisque nous débattons aujourd'hui, certes, du référendum, de son opportunité et des modalités de son organisation, mais aussi du fond du sujet,

de rappeler la logique de cette privatisation et d'expliquer pourquoi cette opération est nécessaire pour l'entreprise, bénéfique pour notre souveraineté et notre sécurité ainsi que déterminante pour l'économie française. J'aborderai

Si cela a pu être le cas dans le passé, les principaux aéroports européens sont en concurrence aujourd'hui. Ainsi, Aéroports de Paris est concurrencé par Heathrow ou Francfort, ainsi que par les aéroports des pays du Golfe.

l'État ! La frontière continuera à être contrôlée de la même manière. La loi, vous le savez bien, l'a rappelé et a fixé les conditions d'exercice des fonctions régaliennes de l'État qui s'imposent et s'imposeront à Aéroports de Paris, quels que soient ses actionnaires. Il n'y aura évidemment aucune privatisation de la police aux frontières

! Nous privatisons également dans l'intérêt d'Aéroports de Paris. (Nous voulons faire d'ADP un leader mondial de l'aéroportuaire. L'entrée de nouveaux actionnaires permettra d'apporter les compétences, les capitaux nécessaires pour améliorer la qualité de service et accompagner le développement de l'entreprise en France,

en avons tiré toutes les conséquences qui s'imposaient à nous. Le cadre de régulation d'Aéroports de Paris sera plus strict après cette opération qu'avant. Nous apportons cinq types de garanties nouvelles. Premier type de garantie : des garanties de cession et d'exploitation avec un cahier des charges précis, écrit dans la loi et dans un décret. Concernant les garanties de cession, les acheteurs devront remplir des conditions strictes de fonds propres et d'expérience dans le secteur du transport aérien pour participer à la cession, et l'État français ne cédera pas ses participations à un autre État ou à une entreprise sous contrôle étatique. Le Parlement a également fixé dans la loi des garanties très précises sur les modalités d'exploitation. Le cahier des charges comportera des points précis ... Lesquels ? ... sur le respect de l'environnement, la qualité des services et le maintien des emplois. Il comportera des garanties sur la présence de l'État : un commissaire du gouvernement et des dirigeants seront agréés par l'État, dont le directeur de la sécurité d'Aéroports de Paris. C'est évidemment déterminant pour garantir les droits souverains de l'État, la protection des personnes et la sécurité des frontières.

tous les cinq ans, l'État et la société fixeront l'évolution des tarifs en fonction des investissements et de la qualité de service, sous le contrôle d'une autorité de régulation indépendante. Encore une ! En l'absence d'accord, fixera, sur avis conforme de l'autorité de supervision, les grandes orientations stratégiques et les redevances facturées aux compagnies aériennes. L'État aura toujours le dernier mot. Je vous donne un certain nombre de garanties, mais vous les écartez écartez d'un revers de main. Pourtant, elles sont importantes ! Deuxième type de garantie : des garanties de bonne gestion de l'entreprise, avec notamment le principe de la double caisse, qui incite au maintien de coûts compétitifs. Troisième type de garantie des garanties de sécurité, avec un cahier des charges strict, contrôlé et soumis à des sanctions. L'État garde le contrôle total des frontières, madame Cohen, vous le savez bien. Sur la police aux frontières, le contrôle des personnes, le contrôle des biens, les douanes, le contrôle aérien, l'État continuera à tout contrôler. Les sanctions pour irrespect des critères de sécurité seront strictes : elles pourront entraîner des amendes à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires de la compagnie.

pour assurer la qualité de vie des habitants des communes avoisinantes et la cohésion de notre nation. Les parlementaires des communes avoisinant les aéroports du groupe étaient inquiets des conséquences de la privatisation. Ils le sont toujours ! Un certain nombre d'entre vous en ont effectivement fait part. Nous avons donc inscrit les garanties dans la loi pour préserver la qualité de vie des habitants, éviter le bruit et l'augmentation

aussi au travers de la procédure du référendum d'initiative partagée, qui dure, elle, depuis huit mois. Nous respectons évidemment l'expression démocratique. C'est la raison pour laquelle nous avons convenu qu'aucune décision ne serait prise pendant la période de neuf mois de collecte des signatures pour la tenue

Le débat public se poursuit. Depuis l'élaboration de la loi Pacte, à laquelle j'ai contribué en tant que député à l'époque, le Gouvernement n'a eu de cesse d'expliquer ce projet de privatisation- ce que je m'évertue à faire encore aujourd'hui devant vous son intérêt et le cadre dans lequel nous souhaitons la mener. Ça ne fonctionne pas ! Le long débat préparatoire et d'élaboration de la loi Pacte, l'implication des élus de la représentation nationale pendant près d'un an,

ont permis l'expression pleine et entière du Parlement sur ce sujet. Le débat public a été largement mené par les promoteurs du RIP depuis plus de huit mois pour essayer d'obtenir, selon les termes de la Constitution, 4,7 millions de signatures. ! Chacun de nous pourra apprécier le 12 mars prochain, sans en préjuger, le résultat de ce long débat. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé devant vous aujourd'hui, au coeur de ce que nous considérons comme un temps fort démocratique, à savoir le recueil des signatures de ce de ce référendum d'initiative partagée. J'ai voulu vous rappeler l'importance de ce projet à nos yeux, et j'espère que cette intervention aura pu répondre,

je me permettrai de dire qu'ils sont parfois erronés. Nous ne privatisons pas les frontières, il n'y a pas de dérégulation au détriment de l'environnement, des riverains, des usagers ou des compagnies aériennes. Nous voulons seulement- je vous le redis, mesdames, messieurs les sénateurs -valoriser le patrimoine de l'État ... Vous le bradez de l'argent public, tout en investissant dans l'avenir des Français,

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie pour ce débat, pour votre écoute et votre attention.